Cher collègue, bonjour monsieur le Ministre, la séance est donc repris. Nous continuons la discussion du projet de loi d'orientation et de programmation du Ministre de l'Intérieur dans la discussion des articles, nous sommes parvenus aux amendements numéro 108 et 167 rectifié bis tendant à insérer un article additionnel après l'article 8 donc 2 amendements identiques à l'étude Monsieur Bénard Roche l'amendement 108. Merci madame la présidente, la présente loi comporte de nombreuses modifications de la procédure pénale et prévoit, ce qui est annoncé comme renforcement de la filière investigations nous pensons de notre côté, que cela doit s'accompagner d'un renforcement des droits de la défense dès ce stade, ce que nous avions déjà porté d'ailleurs par un amendement dans la loi sur la confiance dans l'institution judiciaire comme ne manquera pas de le relever le rapporteur Daubresse cela répond aussi a besoin de confiance avec les forces de l'ordre, l'article actuellement rédigée dans le code de procédure pénale permet au procureur de donner des éléments de dossier mais ne consacrent pas le droit pour les mises en cause et leurs avocats du demander le dossier même expurgé de tous les éléments présentant un risque de porter atteinte à l'efficacité des investigations, à ce stade de l'enquête aussi nous demande, or nous souhaitons renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l'enquête préliminaire en donnant l'accès au dossier au suspect à son avocat dès le stade de la garde à vue, l'étude d'impact du PGA elle confiance dans l'institution républicaine rappeler que dans la plupart des pays européens parmi les droits les plus fréquemment confiés à la personne au cours de l'enquête, figure le droit d'accès au dossier, le plus souvent au cours de la garde à vue et le droit de demander des actes d'enquête ou de participer à des actes d'enquête et d'être informé de ses droits, c'est un amendement qui est travaillé avec le CNPF.

mon amendement va dans le sens de celui qui devient, de vous êtes présenté qui vise à renforcer les droits de la défense, effectivement, l'article 77 de actuelles du code de procédure pénale, limite les le droit à l'accès au dossier pour la partie civile ou plaignants et donne à l'opposé, le pouvoir au Parc au Parc pas au Parc, si, si, au parquet de de son côté pouvoir offrir la possibilité d'un accès au dossier, il paraîtrait plus logique dans ce contexte de consacrer un droit d'accès au dossier pour le plaignant dès le moment de la plainte que de le limiter dans ces proportions, et c'est un petit peu ce que souhaiterait aujourd'hui les avocats, c'est-à-dire pouvoir accéder au tout début de la procédure et dès la clôture de l'enquête aux éléments du dossier qui peuvent lui permettent de préparer sa défense. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur, votre avis. Oui merci madame la présidente, monsieur le Ministre, chers collègues, l'amendement de nos collègues proposent qu'est présentée à deux à 2 reprises, de renforcer les droits de la défense en permettant au suspect et à son avocat d'avoir accès au dossier de la procédure dès le stade de la garde à vue ou de l'audition libre la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire du 22 décembre 2021 qui est relativement récente à renforcer le contradictoire dans le cas de l'enquête préliminaire en permettant à la personne mise en cause d'avoir accès dans certaines conditions au dossier de la procédure, le législateur a cependant veiller à préserver un équilibre entre les droits de la défense et l'efficacité de l'enquête, notamment dans son déroulement, il ne nous paraît pas justifié de rouvrir le débat et de permettre en cause cet équilibre si peu de temps après l'adoption de la dernière réforme et alors que nos concitoyens attendent de la police et de la justice, plus d'efficacité dans les dunes, Lucida sur des affaires, notre avis est donc défavorable. Le ministre ma ma vie parfait je mets donc aux voix avec 2 avis défavorables qui vote pour.

je vais présenter cinq amendements dont je voudrais tout de suite lever un malentendu possible : il s'agit pas de mesures de protection animale, bien évidemment, mais il s'agit de protéger les victimes, il s'agit de prévenir, de dépister et de répondre le mieux possible, au fait, violences intrafamiliales ces cinq amendements sont pas l'objet d'un avis d'une opinion ou d'une thèse ils sont inspiré par un fait établi par des études scientifiques statistiques qui indique qu'il a un très fort lien entre les violences exercées envers un animal domestique dans le foyer et les violences exercées à l'égard de l'épouse ou des enfants, en tout cas du conjoint et des enfants, ce lien statistique il apparaît dans de nombreuses études internationales, vous trouverez quelques références, je peux pas vous infliger de bibliographie maintenant et vous trouvez des des références sur les les exposés des motifs des 5 amendements que je vous ai proposé l'animal est en effet un révélateur de du climat de violence intrafamiliale est l'objet de ces amendements, c'est de prendre cela en compte, mais l'animal est aussi un moyen de pression qui va permettre à l'auteur des violences de mettre de la pression et et d'exercer des menaces sur les personnes elles-mêmes victimes de violences pour qu'elle ne dénonce pas assez fait et qu'elle ne quitte pas le foyer donc animal révélateur animal moyen de pression ces amendements ont été travailler bien sûr avec des professionnels confrontés à ces questions régulièrement et notamment des magistrats, enfin 50 % des ménages ont un chien ou un chat, ce qui fait que, ils sont nombreux à être concernés quand les cas de violence, le premier amendement donc le dix en fait vise à considérer que les sévices graves, les actes de cruauté et les atteintes sexuelles sur animal de compagnie sont des violences psychologiques pour la victime, donc reconnaissance en termes de violence psychologique afin que ce statut de victimes puissent être reconnues et que s'y attache évidemment tous les éléments de prévention prévues Merci, monsieur le rapporteur, votre avis sur ces différents amendements je ne reprendrai pas la parole, pardon, c'est cher collègue, vous avez défendu l'ensemble de vos amendements. Ah, le 1er d'accord n'est pas elle compris. Comme ils sont pas en discussion commune, on va les prendre un par un, même s'il y en a trois dans le code pénal et de dans le code civil de manière de manière liminaire et et je ça fera écho au débat de ce matin, nous ne souhaitons pas à l'échelle de ce texte de loi. Intervenir sur des domaines qui n'étaient pas initialement dans le périmètre, alors ils ont pas été déclarés il ressort-t-il au titre de l'article 45 donc, le débat va, va, va avoir lieu, mais avec mon collègue Marc Philippe Daubresse, nous n'avons mené aucune audition. Des personnes, mon cher collègue que vous évoquez des nous n'avons, nous n'avons entendu aucun scientifique pour la bonne et simple raison que le le le le sujet n'était pas dans le texte initial, donc moi je remets pas en cause le bien-fondé de vos amendements ni le bien-fondé du débat il il doit il doit il doit pouvoir avoir lieu il va avoir lieu, d'une certaine manière, cet après-midi, mais il est important en termes encore une fois, de méthodologie et de capacité de porter les débats au bon niveau que les rapporteurs du texte puisse avoir les éléments sur des éléments aussi importants qui touche au code civil comme au code pénal et que nous que que les rapporteurs puisse proposer à la commission d'avoir un avis qui soit le plus éclairé possible au stade où on discute mon avis de rapporteurs. La vie de mon collègue, co-rapporteur n'est pas suffisamment éclairé pour vous proposer d'avoir un avis vraiment sur le fond, et donc c'est c'est vraiment de de manière assez embarrassé que nous nous sommes résolus à rendre sur ce 1er

c'est de faire figurer des mentions relatives aux animaux de exactement dans les mêmes articles que vis-à-vis des victimes que nous sommes censés protéger oui entame de de de symbolique et de présentation l'pas, nous n'avons pas eu de débat préalable et pas d'audition, j'attire votre attention, mon cher collègue, sur le fait qu'il faudrait peut-être imaginer un dispositif spécifique, plutôt que quelque chose qui vient dans les articles du code civil comme du code pénal qui soit vraiment se où on parle spécifiquement des victimes, qui sont des personnes humaines. Merci, monsieur le rapporteur, pour mon information, vous aurez le même argumentaire sur les cinq amendements. Oui, j'ai envie d'avoir le même moment avant argumentaire sur les les cinq à un moment on va, on va demander notre collègue Bazin de les retirer et à défaut sera un avis défavorable. Très bien monsieur le Ministre.

la capacité qu'ont les auteurs de violences conjugales à s'en prendre, comme l'a dit tout à l'heure, Madame la Ministre, Rossignol aux animaux de compagnie, ainsi soit faire des sévices graves envers ces animaux soit et c'est cumulatif attaquer psychologiquement très sérieusement la personne qu'on a en face de soi et qu'on veut, soit garder pour soi, soit se venger, je mets des guillemets sur elle, donc je comprends très bien ce que vous souhaitez et comment on peut améliorer les choses, puisque cela a été dit par Madame la ministre Roselyne aussi c'est très empirique, la façon dont on gère les les violences intrafamiliales et on découvre à chaque fois, effectivement, un certain nombre de cas de plus en plus importants, notamment parmi les violences intrafamiliales qui se qui se déroulent dans les catégories d'État c'est plus populaire de la population, alors là où on a une difficulté indépendamment monsieur le rapporteur, a évoqué le fait que ce n'était pas dans le texte initial et que ils arrivent en séance et qu'effectivement c'est par ailleurs une des dispositions, je vous renvoie le même argument de monsieur le garde des Sceaux je voudrais pas que ceux qui nous écoutent, crois que lorsqu'il y a des sévices graves envers les animaux, cela n'est pas réprimée, c'est réprimé évidemment dans le code pénal et dans ce il y a des violences psychologiques, ce n'est pas réprimée, c'est également présent dans le code pénal, mais ce que j'ai bien compris, c'est que vous souhaitiez en faire une discrimination positive pour bien le souligner afin que dans les ordonnances de protection dans la condamnation des personnes, on puisse voir les choses de façon aggravé, mettre en en en en avant ce phénomène tout particulier, il me semble en effet que le rapporteur n'a pas tout à fait tort lorsqu'il dit qu'il ne faut pas le mettre de manière parallèle, les personnes et notamment les victimes, et singulièrement les femmes et les animaux qui sont parfois les victimes aussi, mais qui ne relèvent pas évidemment dans le droit français tels qu'il est écrit : jusqu'à présent des mêmes évidemment protection que les personnes humaines donc tout en ayant bien conscience de votre sujet qui a été évoqué aussi pas votre collègue, ce matin, proposé de pouvoir les retirer également pour qu'on puisse y travailler notamment lorsque le garde des Sceaux va présenter, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui depuis plusieurs heures sur les avancées annoncées par exemple la première ministre ou sur les violences intrafamiliales, je pense à la justice spécialisée mais aussi au rapport que rendra votre collègue sénatorial qui pourrait éventuellement reprendre aussi des dispositions qui concernent les animaux domestiques dans le cas des des séparations dans le cadre des violences commises au sein du couple, donc un avis défavorable à préretraite. Très bien monsieur Bazin vous retirer. Non, alors, explications de vote de Madame Rossignol. Merci madame la présidente, je j'ai eu l'occasion ce matin monsieur médecin je sais pas si vous étiez dans l'hémicycle comme je vois pas bien d'évoquer ces amendements à l'appui de mes démonstrations sur l'ordonnance de protection. Et je voulais dire que en ce qui me concerne, je voterai cet amendement et faute, il faut bien comprendre de quoi il s'agit, il ne s'agit pas de faire rentrer la condition animale dans le code civil, il s'agit de mieux définir ce que sont les violences psychologiques, c'est ce que c'est le cas du premier amendement et on sait bien suffit de lire les journaux, de s'intéresser un petit peu différents sujets aujourd'hui pour identifier que en ce qui concerne les violences psychologiques, nous sommes encore dans des définitions soit psychologiques soit jurisprudentielle mais que un certain nombre d'éléments ne sont pas encore clairement identifiées comme relevant des violences psychologiques, ce que dit l'amendement sous votre contrôle, chers collègues, c'est que le fait d'exercer des violences sur un animal dans une, est une violence psychologique exercée, non pas sur l'animal mais sur les autres membres du foyer, c'est-à-dire le plus souvent la femme et les enfants et Monsieur le Ministre, dans un domaine que vous connaissez bien, qui est la lutte contre la radicalisation et le terrorisme, nous savons qu'il existe des signaux faibles. Voilà, ce concept de signaux faibles, on ne connaît pour la radicalisation, hé bien la violence contre les animaux est également un signal faible en matière de violences intrafamiliales, c'est pour ça que le l'idée et le le fil conducteur des amendements de notre collègue Bazin et juste, et l'amendement hé bien placé, je dirai un mot tout à l'heure parce qu'à cinq amendements, j'aurai l'occasion de m'exprimer une deuxième fois sur un petit problème quand même sur notre capacité d'amender en séance qui commence à poser un petit problème parce que, apparemment, c'est plus possible

qui viennent d'être d'ailleurs bien illustré par notre collègue Rossignol, qui a manifestement bien compris en effet que cet amendement se borne à reconnaître le fait que des violences physiques sur un animal du foyer représentent des violences psychologiques pour les autres, pour les personnes du foyer, évidemment, c'est ça, et seulement ça l'objet de l'amendement et il me semble que c'est relativement évident et que ça a quand même une portée importante en permettant de considérer les enfants ou le le conjoint comme des victimes de ces violences psychologiques et ça donne un cadre un peu plus solide en effet au juge qui veut apprécier tout cela, par ailleurs, ce matin, j'ai bien entendu que il peut être difficile pour le rapporteur, et pour la commission de d'exprimer une opinion sur un sujet quand qui n'a pas été expertisée à fond et je peux comprendre ça cependant ce matin que ça va apporter un amendement qui ont pour beaucoup plus de complications d'appréciation que ce que je vous propose là et il a été décidé de lui faire un sort quand même relativement favorable puisque il va aller dans la navette, ce que j'ai compris. rapport alors. Mais, mais il a été voté, donc ça permettra quand même d'avoir le débat, ensuite on verra bien quel sort sera réservé à ses amendements, mais l'essentiel c'est que on puisse entendent dans cette assemblée, qui a un sujet important autour des violences qui ont lieu dans le foyer sur les animaux et que c'est uniquement 100 absolument mettre sur le même plan l'homme et l'animal, ce que ne fait aucun de ces amendements, c'est simplement prendre ce fait en considération pour progresser dans la prévention et le traitement de ces violences. Merci, chers collègues, monsieur le rapporteur. Oui, parce qu'il faut, il faut quand même maintenant venir pardon, on a dit ce matin que la commission des lois, été attentive à la rédaction du code pénal et à la rédaction du droit en général, on va, si cet amendement était adopté, modifier le code pénal. Je le dis dans un loi d'orientation de programmation de ministère de l'Intérieur et malgré les, les, les observations qui ont été les miennes, puis celle du ministre, c'est-à-dire que on on est on est on est vraiment, alors que la commission des lois n'a pas pu auditionner alors que la commission des lois a débattu de ce sujet-là et les mêmes observations ont été formulés devant les collègues. l'article que vous voulez modifier mon cher collègue que vous voulez compléter, dis donc, ça, c'est l'article 222 14 tiré trois les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées, quelle que soit leur nature, y compris lorsqu'il s'agit de violences psychologiques et ensuite vous introduisez le dispositif que vous avez prévu, c'est-à-dire que vous allez faire, à la suite d'un d'une tête de de de chapitres qui est général. Faire un cas particulier. Dans lequel vous évoquez, pardon de le dire, dans le même article les personnes humaines, victimes de violences et évoqué la situation des animaux eux-mêmes victimes de violences pour en faire un facteur aggravant, enfin si je vous je vous alerte sur le fait que cet élément figurant dans le même article, moi, me pose un problème de fond et que nous, je n'ai pas pu mener aucune audition et ne je n'ai pas pu entendre les scientifiques dont vous avez pas dont vous avez parlé tout à l'heure, ça me pose un vrai problème de méthode hein et et de et de porter, y compris dans la navette une modification du code pénal sur ces sujets-là, pardon, d'en faire un un peu un un élément de gravité mais pour pour le la, le, le, le bon déroulement des travaux du Sénat et le sérieux de la commission des lois, ça me pose une vraie difficulté que j'ai déjà évoqué à 2 reprises au sein des travaux de la commission et que je tiens à évoquer ici en séance publique.

qui vote pour. Qui s'abstient, il n'est pas adopté.

je veux même pro vous proposez de de soutenir le 11 et le 12 en même temps, puisqu'en fait, le douze est un amendement de repli, il s'agit en fait dans l'amendement numéro 11 de proposer que soit constitutif de harcèlement. Les propos ou comportements à l'encontre d'un animal de compagnie détenues au sein du foyer ont pour objet ou pour effet de créer à l'encontre du conjoint du partenaire lié par pacte civil de solidarité ou du concubin, une situation intimidante, hostile ou offensante, il s'agit en fait de reconnaître le rôle des menaces sur l'animal comme constitutifs du délit de harcèlement et dans le l'amendement suivant amendement de repli, il s'agit de considérer la que l'infraction est constituée l'seulement quand ces comportements mettent en danger l'animal. Merci, monsieur le rapporteur, donc défavorable, vous êtes déjà exprimé sur le sujet, me semble-t-il, monsieur le président de la commission, vous vouliez dire. Ah je je ne voudrais bien et sur le fond, madame la madame la présidente, si vous le permettez, cet amendement pose un un problème important puisqu'il aboutirait à ce que le délit de harcèlement moral du conjoint soit plus facile à constater, lorsque le harcèlement vise un animal que lorsque le ce harcèlement vise le conjoint lui- même, je m'explique : pour que le délit de harcèlement moral soit constitué, il faut que le conjoint soit victime de propos de comportements répétés ayant pour effet ou pour objet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, vous le voyez, les conditions à réunir sont strict. Avec l'amendement que vous proposez, mon cher collègue, le harcèlement de l'animal, constituerait un délit s'ils créent simplement une situation intimidante, hostile ou offensante pour le conjoint harcelée un animal serait ainsi plus facilement punissable que harceler son épouse ce qui nous paraît une cohérence tout à fait relative, l'avis est défavorable. Monsieur le Ministre, même avis défavorable, ce président de la commission, vous vouliez ajouter quelque chose. Alourdir le débat mais je voudrais dire à notre collègue Bazin que l'amendement précédent n'a pas été adopté, je ne sais pas quel sera le destin des autres et l'engagement que je peux prendre dans l'occasion de cette séance et le fait que la commission des lois aillent dans un débat et étudie la situation que vous avez, nous sommes à peu près tous d'accord sur le constat que vous faites et que vous dénoncez, en réalité, il y a pas de difficulté là-dessus la question tout le monde l'a bien compris, c'est une question de de forme et et juridique alors la commission des lois, ne fait pas du droit pour faire simplement du droit, le droit n'est qu'un moyen, mais si on veut que on, on arrive à quelque chose qui fonctionne et qui puisse satisfaire la demande qui est la vôtre, moi je m'engage aujourd'hui, devant vous, devant les collègues à faire un travail à engager un travail au sein de la commission des lois, voilà, c'est ce que je voulais vous dire simplement. Monsieur Bazin pour explication Bush. Merci madame présidente, monsieur le Ministre, je voulais remercier le le président de la Commission pour cet engagement que je reçois avec plaisir et très volontiers, donc je lui fais totalement crédit juste une observation sur ce sur cet amendement, là j'ai entendu les observations du rapporteur sur les adjectifs qui qualifient donc les propos. Et qui font en effet un problème que je reconnaîtrai volontiers on monte devra retravailler ça, donc je vais retirer cet amendement là les autres, on va quand même les présenter encore une fois, pour que tout le monde des ententes, cependant je fais observer au rapporteur, que pour le coup, c'est lui qui met sur le même plan le l'homme et l'animal, puisqu'on ne concerne on ne considère le harcèlement on considère le harcèlement de la personne à travers les les sévices ou actes inappropriés sur l'animal, l'animal lui il est qu'un révélateur : il n'est pas du tout au niveau de la personne, il faudra qu'on conserve tout ça dans les textes tels qu'on les envisagera donc merci, merci pour vos propos, monsieur le président, et puis présidente je je retire celui-là. Et de vous avez présenté les 2 11. Oui, oui, puisque c'était un amendement de repli là les mêmes observations. Fais nous passons donc à l'amendement numéro un monsieur Bazin. Il vous en reste deux il y a le A et le deux. Allez-y, allez-y. Alors sur l'amendement numéro un, là on est au au code civil, il s'agit de prendre en compte les animaux de compagnie détenues au sein du foyer, les violences, qui sont plutôt commises à leur égard pour permettre les conditions de de les considérer, dans les conditions de déclenchement des ordonnances de protection des victimes de violences intrafamiliales, en effet, cette ordonnance de protection du juge civil n'est pas conditionner l'existence d'une plainte pénale et comme je l'ai dit tout à l'heure un comportement violent s'applique de façon globale, à ceux qui les entourent, d'autant plus qu'ils sont aisément vulnérables. Cette violence unique qui peut exister au au sein d'un foyer mal connue en France et les plus reconnus à l'étranger et les études dont je parlais tout à l'heure sont largement des études anglo-saxonnes, mais pas seulement, dans un contexte d'augmentation de violences conjugales depuis plusieurs années, en dépit des mesures déployées depuis le Grenelle éponyme, il serait incompréhensible de se priver d'un tel indicateurs dans la validation dont la validation dans nos ports. Aucun effet délétère, il s'agit donc essentiellement de permettre aux juges de prendre en compte ces violences sur l'animal par un des conjoints pour prononcer une une ordonnance de de protection, c'est donc là l'utilisation de l'animal comme un révélateur du climat de violence. Merci, monsieur le rapporteur, avis défavorable. Oui, madame la présidente, le la vie sera toujours défavorable mais mais quand vous lisez le le dispositif législatif monsieur monsieur le mon cher collègue à l'article 515 tiré 9 du code civil après le mot enfant au pluriel sont insérés les mots ou les animaux de compagnie détenues au sein du foyer, vous imaginez la réaction qui peut te la mienne quand je lis ça, je comprends que vous dites que les animaux sont un révélateur que de manière statistique et empirique, quand il y a de la vous dire sur l'animal, souvent on peut constater qu'il y a ou qu'il peut y avoir de la de la violence sur conjoint néanmoins faut c'est pas moi qui met sur le même plan, parce que quand vous mettez un où entre les enfants où ça ça peut créer une une réaction, une une une interrogation, en tout cas de, de, de notre part, donc, la vie est est toujours défavorable, il est d'autant plus que il sera par cohérence avec les arguments que j'ai pu développer ce matin à l'égard des amendements de Madame Rossignol. L'ordonnance de protection est un dispositif complexe sur lequel nous avons décidé au sein de la commission des lois, de ne pas intervenir à l'échelle de ce texte là, donc nous avons ce matin eu été suivi majoritairement par les collègues dans cette assemblée pour ne pas modifier l'ordonnance de protection, il y a des travaux Chandler vers rien, qui sont en cours, il y a des personnes à entendre le sujet mérite d'être mis sur la table, c'est une évidence, mais l'ordonnance de protection éteint n'objet juridique suffisamment sensible pour qu'on y touche du non pas d'une main tremblante mais qu'on est con con la réforme clairement mais une fois qu'on aura à mener des travaux qui permettront à chacun de s'exprimer et avec des travaux qui seront éclairés, mais vous voyez quand vous voyez le le dispositif que vous proposez dans le dans, je suis très interrogatifs quand même, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un dispositif propre séparé du disposer des dispositifs existants. Monsieur le rapporteur, monsieur le Ministre, même avis défavorable. le signal pour explication de vote ah et Arnaud Bazin vous vouliez le retirer non. J'ai tenté après moi je vais également soutenir ces amendements comment dire les choses, délicatement, pour ne pas froisser les collègues si sensible et qui sont toujours très, très affecté par menace ou mes chantage mais ce qui, mes chers collègues, ce qu'a de plus sensible, c'est pas l'idée qu'on peut se faire de ce que produirait l'effet de l'introduction dans le code civil de cette disposition, ce qui est plus sensible, c'est la somme des violences commises dans les foyers, contre les femmes et des enfants. j'ai utilisé vos amendements ce matin justement sur l'ordonnance de protection à propos, la question des menaces, par exemple, j'ai pris d'exemple quand un homme dit je vais tuer ton chat ou ton chien et on veut évoluer les animaux tu les reverras jamais, c'est une menace qui devrait justifier une ordonnance de protection, c'est pour ça que vos amendements, j'en suis absolument convaincu sont nécessaires et je n'ai aucun problème pour aller expliquer ça à l'extérieur, l'effet que ça va faire, mais les gens comprennent très bien quand on leur dit : quand on leur explique que les violences sur animaux sont une violence psychologique sur tout le foyer et en et de surcroît un risque accru de violence sur les membres du foyer, par ailleurs, je voudrais quand même dire à mes collègues de la commission des lois, quelque chose qui m'échappe un peu, parce que vous avez des amendements depuis 8 jours, comme moi, puisqu'ils ont été déposés en commission par notre collègue Bazin, ils m'ont été transmis à l'issue de la commission pour avis, j'ai eu le temps de les étudier pendant huit jours vous dites que vous n'avez pas pour votre part pu les examiner les, les, les, les expertiser mais ça pose un problème, ça veut dire qu'en fait tout amendements déposés en commission et qui n'est pas adopté par la commission ou qui viendrait même en séance ne peut pas être directement et et de au motif que la commission des lois, ne pourrait pas l'avoir précédemment expertiser, valider sa porte légèrement atteinte quand même au droit d'amendement que chaque parlementaire, à qui est égal sur tous les textes, quelle que soit la commission dont on est membre. monsieur Bazin vous avez demandé la parole pour une explication de vote. Merci madame la présidente, ce ministre juste 2 observations, suite aux propos de monsieur le rapporteur, tout d'abord, c'est pas parce qu'on met dans une même phrase. phrase. 2 mots qu'on met nécessairement les choses qui sont derrière, sur le même plan, sinon je crois qu'on peut faire un peu d'expertise, ça va quand même être compliqué de faire tenir tous les textes donc premières observations, deuxièmement, si on met cette disposition dans un autre texte, je ne vois pas comment on peut le faire puisque le coeur de la mesure, c'est de mettre la cet élément de révélateur de prise en compte des maltraitances sur l'animal domestique pour prendre une ordonnance de protection pourrait-on le mettre ailleurs que dans leur danse dans les textes qui concernent l'ordonnance de protection là je j'ai du mal à suivre sur les précédents, peut-être y a-t-il des solutions, on verra, mais la dessus, j'ai un peu de mal à suivre, c'est pourquoi je pars cohérence c'est par conviction, je je maintiens l'amendement et en tout cas j'essaie de faire vivre ce sujet au sein de notre assemblée. pardon de vous contredire, mon cher collègue, mais le le le le texte, c'est lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation par l'ancien conjoint un partenaire lié par un Pacs ou un ancien concubin, y compris sur ce qui n'a jamais eu de cohabitation mettent en danger. La personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants ou.

un ou plusieurs enfants ou des animaux de compagnie en en français, non pas en droit mais en français vous êtes sur le même plan, c'est pour ça que moi je suis, je suis très très réservé sur vos amendements, c'est le moins qu'on puisse dire hé et Madame Madame on n'a jamais interdit à quelle a aucun de nos collègues de déposer des amendements, il y a les amendements qui ont été qui ont reçu des avis favorables sur tous les bancs de cet hémicycle, simplement on a estimé que, il y avait une un Champ qui est celui de l'ordonnance de protection pour lequel nous n'avions pas mener les auditions pour lesquels nous n'avions pas le temps de les mener depuis une semaine pour ouvrir ce Champ là et donc ça a été un choix de ne pas le faire, sachant qu'en plus, je le répète, d'autres travaux parlementaires sont actuellement en cours. Je mets donc on voit cet amendement madame de rien. j'entends bien, et c'est évident qu'un animal de compagnie, peut être un objet transactionnel et et que on en en s'attaquant à l'animal, on s'attaque directement à son propriétaire et j'imagine bien que si mon mari se tenait ma chienne du 5ème étage en disant : si tu es pas gentille, je la je la chienne, je serai à mon avis très gentille, pour récupérer la chienne, c'est la première fois, pour autant qu'on parle du de, de, de cet objet et mais je l'entends et donc je pense que je j'entends bien aussi qu'il a probablement un problème d'écriture à travailler, mais franchement j'entends, j'entends ça très bien, et donc je vous promets que ça fait partie de la liste que je mets des choses à étudier par rapport aux violences intrafamiliales. Merci, je mets donc aux voix cet amendement avec 2 amis défavorable qui vote pour. Qui vote contre.

non pas parce qu'on les considère à l'égal des personnes qui sont dans le foyer, mais parce que quelques études et notamment une nous dit que dans près de 50 % des cas où la l'épouse, c'est que quand même le cas le plus fréquent, a dû quitter le foyer, elle a retardé son départ à cause du sort de l'animal domestique, donc c'est le moyen de pression dont je parlais tout à l'heure donc, en donnant la possibilité au juge de statuer sur la garde pas sur la propriété, c'est un autre sujet, mais en urgence sur la garde, on lui permettant à au conjoint de partir avec l'animal pour le soustraire aux violences qui sont éventuellement évoquée par le conjoint pervers qui cherche à maîtriser la situation, garder le contrôle, hé bien on permet à la jointe de se mettre en sécurité plus rapidement dans 50 % des cas il elle est retardée, voilà, c'est l'objet de cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la présidente de l'avis sera défavorable, je rappelle à notre collègue que normalement le la meilleure des solutions, c'est l'éviction du conjoint violent plutôt que le départ de la personne victime de violences. Monsieur le Ministre votre avis.

Nous raisonnons tous tous services de police et de gendarmerie autorité judiciaire et du locaux qui mettent à disposition un certain nombre de logements, bref pour dire que nous devons sortir la dame puisqu'il s'agit très souvent d'une dame, ça peut être parfois monsieur mais très, très souvent, une dame de son lieu d'habitation. Et vous parlez des animaux domestiques, je pourrais aussi parler des cas que j'ai connu quand j'étais maire de dame qui était par exemple l'assistante maternelle qui avait l'agrément du conseil départemental pour exercer leur métier dans l'appartement ou la maison elle et et qui ne pouvait pas partir ou retarder le départ du fait de son conjoint violent parce qu'elle avait perdre son métier en même temps qu'elle allait perdre son couple, pardon de le dire comme ça, donc je pense qu'il y a plein de dispositions qui permet de réfléchir, je crois à une généralisation ou au moins en tout cas à une possibilité de cinquante cinquante, on va dire ça comme ça, de qu'est-ce qui est le plus important est-ce que c'est d'éloigner le conjoint violent ou d'éloigner la dame, ben personne en tout cas qui être victimes de cette violence, ça peut être des animaux, vous l'avez tout à fait bien dit ça peut être son métier, ça peut être des objets auxquels elle tient, ça peut être plein de son voisinage, ça peut être sa maman qui habite à côté et voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles il y a des freins ah il y a aussi des raisons pour lesquelles il n'y a pas assez de logements d'urgence et dangereux continue d'urgence il y a aussi un tabou dans la société qui est d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait du conjoint violent notamment quelles quelles sanctions on lui mais indépendamment des sanctions pénales, bien évidemment, tout, je pense que dans vos futurs réflexion, je me permets de dire à madame la sénatrice qui qui s'occupe de ce de cette mission, mais à d'autres, la question du lieu et qui doit rester dans le lieu est très importante, mais comment on fait appliquer le fait que personne ne revienne dans ce lieu, ce qui est le problème de l'éloignement des des des conjoints des conjoints violents par exemple, il m'a semblé moi dans ma vie d'élue locale, que c'était le manque d'habitats spécifiques pour accueillir les conjoints violents qui était la cause principale du fait qu'on ne les éloigner pas et non pas parce que la loi ne prévoyait pas, mais parce que dans le monde réel, comme vous l'avez dit, à travers les paroles de l'hémicycle, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, donc moi je prend bien en compte évidemment la question des animaux domestiques, je ne les sous-estime absolument pas, on pourrait imaginer plein d'autres cas il y a pas d'autres cas, pour lequel on éloigne pas le conjoint violent mais on éloigne l'affaire. Ce qui est la victime et du coup elle retarde parfois son départ pour plein de raisons qui relève notamment, sera un moment et plein d'autres sujets donc défavorable sur le l'amendement parce qu'on a dit qu'on travaillé ça pour plus tard, si je peux me permet d'être grossier ainsi mais je trouve que c'est une très bonne question. Merci, Monsieur le Ministre Monsieur Bazin pour explication de vote. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, moi je j'entends bien tout ce qui est ce qui a été dit, là, mais je voudrais surtout pas qu'on reste sur l'idée que on s'est préoccupé du sort des animaux domestiques dans ce débat, on s'est préoccupé du sort des personnes victimes de violences et on s'est interrogé sur la pertinence de prendre des mesures de considérer que d'animaux domestiques sont des révélateurs de ces violences, ils doivent être pris en compte et prendre des mesures pour faciliter la protection donc des personnes à travers les animaux domestiques, ça c'est le le 1er point que je voulais souligner et puis sur l'éloignement du conjoint, on est tous d'accord que c'est le violon qui doit être en éloigner dans la mesure du possible, en priorité, il n'empêche que même dans ce cas, le rôle là il y a un sujet sur la garde le la détention de l'animal qui peut être sujet à hein, donc des menaces ou même à déjà à des violences perpétrées,

Ces amendements n'ont pas été accepté non, celui-là ne le saura-t-il pas aussi, mais il était indispensable que toutes ces matières là soient maintenant retravailler comme l'engagement, on a été pris. Merci Madame Rossignol pour explication de vote. c'est plus pour les réseaux sociaux que pour nous même, nous n'avons pas cherché à créer une ordonnance de protection pour les animaux, je tiens à préciser, à la fin de ce débat, l'ordonnance de protection et toujours pour la femme, enfin pour le conjoint qui qui la demande, ça c'est la la première remarque Elle protège également les enfants et Monsieur notre collègue Bazin hé bien expliqué le à quel point les animaux pouvaient être un objet soit transaction de de chantage noble un un objet de de souffrance et de pression, mais juste une chose : dans les divorces on statue sur les animaux, sur qui gardent les animaux domestiques, donc c'est pas absurde de statuer aussi sur leur demande dans l'ordonnance de protection, mais j'ai bien compris que c'est pas aujourd'hui qu'on va réformer l'ordonnance de protection, j'espère que ça mettra pas trop longtemps quand même pour venir, j'ai eu l'occasion de le dire ce matin et puis enfin sur l'histoire, j'entends souvent le le principe c'est l'éviction du conjoint violent et, quand il a passé 48 heures en garde à vue, qui est le mieux qu'on puisse faire ou en cellule de dégrisement aussi et qu'après il ressort et que là

avec anonymisation de mon lieu de résidence qui n'est pas prévu non plus par l'ordonnance de protection et qui fait partie de mes amendements et des sujets que j'espère traiter. Oui, mais puisque non, non, enfin, on peut toujours discuter non, en tout cas c'est pas, c'est pas avec moi que vous aurez ce problème-là, non, j'en profite puisqu'on parle de ce débat très important et qu'on parle de choses qui dans le monde réel, fait que on a du mal à. Il y a aussi une difficulté pour les bailleurs sociaux, parce que souvent on peut trouver un logement social à la personne, il faut que l'on prévoit le fait que lorsqu'on est propriétaire de sa maison, de son appartement et ça arrive, y compris dans la classe populaire là où on a des difficultés où s'accumulent les difficultés sociales, on ne peut pas trouver un logement social à une personne, même lorsqu'elle est victime de violences conjugales, si vous êtes propriétaire d'un logement, et ça c'est quelque chose je crois qu'il énerve à peu près tous les élus de France, il faut avoir été maire ou en tout cas, élu local très implanté pour le savoir, il faut que le Parlement, je le regarde, parce que là c'est pas du tout ma compétence mais je le dis que j'ai le bonheur de pouvoir parler à ce micro, ce que ne font pas l'immense majorité des citoyens français, donc je me permets de le dire. Ici, bien évidemment, il faut absolument qu'on trouve des moyens dans les textes législatifs qui touchent le logement ou qui touche peut être la justice quand on parlera des violences conjugales, on doit pouvoir donner un logement social à une dame ou un monsieur qui correspond à la vie familiale et, notamment, à la vie des du nombre des enfants qu'on doit avoir de manière expresse sans attendre un jugement définitif qui condamne l'auteur de cette personne parce qu'on met ça met parfois du temps et surtout sans avoir besoin de demander la vente d'un immeuble d'un bien qui met toujours du temps et dont le la personne qui est responsable des violences dans le couple utilise pour le coup en violences psychologique le divorce et la vente du bien pour pouvoir refaire sa vie. Quand on est parti du cycle du retour de la victime envers son agresseur, donc je veux dire aussi signal mais je sais qu'elle le sait, l'un des freins sur le fait on arrive pas à régler ce problème aussi, c'est que notre politique de logement et tout à fait incongru par rapport à la politique, on essaie de mettre en place, ce sont des violences intraconjugales. Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Qui vote contre.

Merci qui vote contre.

Nous passons à l'article 9 avec 4 amendements identiques de suppression le 35 4 amendements. Monsieur l'amendement numéro 35. Oui, madame la présidente, je vais déposer le 1er amendement de de suppression. L'article 9 s'inscrit dans le chapitre renforcer la filière investigations et et dans ce chapitre, renforcer la filière investigation s'est renforcé qui nous inquiète, alors l'amendement de suppression était un peu radical, mais il vient traduire quand même une une très profonde inquiétude que nous ne sommes pas les seuls à manifester parce qu'il nous semble quand même que, assurer la qualité des des actes de police judiciaire nécessaire au au déroulement et et au bon déroulement et à la qualité des enquêtes, c'est essentiel, alors vous vous souhaitez au travers de de cet article 9, tirer les conséquences de la réforme de la formation d'OPJ en intégrant dans la formation initiale des gendarmes et des gardiens de la paix, la suppression de la carence de 3 années et il nous semble que. Rechercher le nombre, l'effectif et vous l'avez exprimèrent vous êtes vous êtes exprimé très longuement hein sur sur ce sujet le le besoin de de nourrir les filières investigations, ce n'est pas de nature forcément à renforcer ses ses filières, en réduisant les exigences de pratique et d'expérience requises pour devenir OPJ il nous sommes qu'on risque réellement d'affecter à terme la qualité des actes peu judiciaire de fragiliser les enquêtes même et de pénaliser ainsi la manifestation de la vérité, la protection des victimes, donc il nous semble que finalement cette accélération de l'entrée dans le métier d'OPJ et peut être de nature à affaiblir la fonction. Merci Monsieur Bénard Roche même amendement numéro 57. Oui je je vais compléter les propos de Jérôme Durain, que je partage totalement : en fait, si cet amendement de suppression donc pour obliger de supposées de s'opposer à la suppression de la durée minimale d'expérience de gendarmes et des policiers deux 3 années pour être habilité en qualité d'OPJ, c'est que nous pensons effectivement que cette mesure va revenir à supprimer de l'expérience au service de l'expérience sur le terrain et à réduire considérablement l'expérience en qualité d'APJ des jeunes recrues, nous ne sommes pas le seul à le dire, vous, vous le savez d'autre aussi bien du côté de la police, que du côté des avocats l'ont déjà dit, et ont exprimé des inquiétudes sur l'amoindrissement inéluctable des compétences et de la qualité des futurs OPJ avec une telle réforme de leur formation, vous savez que les OPJ, un certain nombre de pouvoirs coercitifs des placements en garde à vue des demandes de réquisition des deux mois de perquisitions des visites domiciliaires, ce qui suppose effectivement de leur dispenser une formation de la meilleure qualité possible et la condition d'ancienneté donc deux 3 années en tant qu'PJ nous apparaît également primordiale et nécessaire pour acquérir expérience et maturité qui sont demandés pour ce type de poste ça consiste en quelque sorte, pour nous, cette réforme a baissé quelque part le niveau d'exigence dans la formation des OPJ et à terme baisser ce niveau d'exigence ne peut que baisser ou porter atteinte à la qualité des enquêtes, c'est pour ça que nous demandons la suppression de cet article. Si Monsieur Favreau amendements identiques. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, chers collègues, je je porte un amendement de suppression comme mais mes 2 collègues, je pense que les arguments qu'ils ont développé, sont parfaitement pertinent, ça rejoint d'ailleurs un petit peu une une vague de de déclassement d'un certain nombre de professions aujourd'hui en France, je ne veux pas citer tous les domaines dans lesquels on peut quelquefois se poser des questions, ça vaut un petit peu pour l'éducation, ça vaut aussi un petit peu dans le monde de la santé et je pense que, effectivement, il est important sur une matière qui est une matière d'une particulière importance pour ceux qui sont concernés, hé bien, il est important que les OPJ garde les compétences qui sont les leurs, actuellement. Merci madame la présidente pour être habilité en qualité d'OPJ, je dois dire. Que mon groupe a auditionné très longuement, bien évidemment, des magistrats, des avocats et y compris des policiers et tout se disent opposés à cet article 9 les éléments, les arguments ont été donnés par mes collègues précédemment et bien évidemment je les rejoins et je confirme donc notre volonté de supprimer cet article. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis. Madame la président de la possibilité pour les policiers et les gendarmes de passer l'examen d'officiers de police judiciaire à l'issue de leur formation initiale se traduit surtout par un enrichissement de cette formation, comme l'ont indiqué le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le niveau de l'élite de l'examen ne changera pas et si les élèves n'ont pas le niveau, ils ne réussiront pas le concours bout de trente où ils ne pourront avoir la qualité de biche d'OPJ qu'au bout de 30 mois de service d'au moins six en tant qu'agent de police judiciaire, il paraît dès lors utile de laisser la chance à cette réforme, qui peut être positif pour toutes les nouvelles recrues mieux former la procédure pénale et pour la police judiciaire, notre avis est défavorable. Merci, monsieur le Ministre, ma ma vie. Oui, mais alors là, je vais prendre un tout petit peu de temps, pas beaucoup mais un tout petit peu de temps parce que je ne comprends pas, Monsieur Durand, vous, surtout qu'il a participé au mauvais la sécurité bon non, je ne voudrais pas vous devez compromettre le sénateur

Que nous avons tous à trouver des officiers de police judiciaire et à faire un code de procédure pénale appliquée et c'est très heureux pour tout le monde correctement de dégrader la formation d'OPJ pour que grosso modo on dégrade la qualité pour avoir la quantité on baisse le taux pour augmenter la base pour parler comme un ancien ministre des Comptes publics. Ce n'est pas du tout l'objet de l'article. Puisque je dis à monsieur le sénateur ben Roche, qui a défendu à peu près cette idée, voilà quelques-uns. Attends, nous ne touchons ni au concours. Ni à la façon dont passeront cours ni au contenu du concours ni à ceux qui préside de concours qui sont les magistrats. Il s'agit et c'est l'objet de l'article d'anticiper pour une partie des gardiens de la paix et des gendarmes de passer ce concours avant une clause qui avait été mise qui consiste à dire : il faut que vous ayez au moins 3 ans d'expérience avant de passer le concours Est ce que les trois ans que l'on passe en tant qu'PJ suffisent pour garantir une certaine expérience. alléger les les compétences du Goncourt, j'aurais tendance à vous dire, mesdames, messieurs les sénateurs aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre des années, on peut faire, disons, de police et être un mauvais procédurier. Et on peut entrer à l'école de police, je les ai pris cet exemple de gens qui ont des licences de droit des master de droit il y a même des avocats qui passe le Goncourt de la police nationale et qui se retrouve donc après avoir fait 12 mois d'école parce que par moments, il faisait mois d'école à attendent 3 ans pour pouvoir passer le concours de PJ bah, excusez-nous, mais ça n'a rien à voir l'Jean tout ça, là, je ne fais rien à l'affaire, comme disait Georges Brassens : quand on n'est pas bonne de PJ, on n'est pas bonne OBJ pour reprendre sa formule, donc il faut. Rester raisonnable et considérer que, il y a plein de gens qui aimeraient rentrer passer des concours de la police et de gendarmerie et peut être même d'ailleurs que c'est ce que vous souhaitez diversifier les profils de gens qui ne veulent pas faire de la sécurité publique, mais réfléchir à la procédure, vous les empêcher de le faire, parce que si demain j'arrête et des 10 intérieur et je me disais tiens j'ai envie de passer un concours de la police nationale, ça peut arriver à chacune et à chacun, rue surtout que j'ai fait sauter la limites d'âge désormais on peut le passer à n'importe quel âge ce concours de la police nationale gendarmerie on pourrait imaginer, je pourrais être peut être être policiers ça ne ça ne veut rien dire en tout cas je passe le concours, on imagine que j'ai réussi, j'ai un peu d'expérience de la vie professionnelle, petite, j'ai notamment été maire de ma commune, donc ce qui me pousse peut être avant, petite expérience d'ailleurs de la police judiciaire, et j'ai un diplôme de droit, bon, je vais vous passer le concours, je l'aurai, j'ai passé ma formation et on dira non. Il faut attendre 3 ans dans un commissariat en tant qu'PJ pour pouvoir éventuellement passer le concours, écoutez, j'ai 40 ans, ça fait encore si je passe le concours, j'en aurai 41 12 mois de formation, ça fait 42, je vais donc dire à ma femme, bon ben attends, bouge pas, je vais passer le pays, dans 3 ans et dans trois ans, je suspends ma vie professionnelle, pardon. Oui, mais en l'occurrence, je suis un homme là j'en suis désolé c'est ça, je peux faire beaucoup de choses pour vous plaire Madame Rossignol, mais je crois que à ce poids de notre discussion, je vais rester dans mon genre, bon, en tout cas, là tout de suite, comme dirait le rapporteur, on n'a pas pu étudier des choses tout de suite donc on fera ça de séance. Or gars, je veux dire à chacune et à chacun trouve ou que je ne ferais pas cet examen parce que je veux dire je vais pas prendre le risque professionnel de changer de voie, il y a plein de gens qui change de voix aujourd'hui. parce que je vais apporter mon expérience dans la police et gendarmerie en disant : voilà, en fait, on ne fait pas confiance, il y a falloir que je suspends de nouveau ma vie professionnelle, ma rémunération pour passer ce concours, donc ça me paraît objectivement des défense hasardeuse, troisièmement, qu'est-ce qu'on a trouvé comme moyen d'atterrissage avec le garde des Sceaux, parce que vous aurez compris que c'était un amendement qui a en commun avec le garde des Sceaux. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme moyen, c'est que vous n'avez pas la qualité d'OPJ immédiatement après l'école. je voulais rappeler et ça fait écho à notre discussion de l'année dernière sur l'allongement de la formation des policiers et des et des gendarmes, puisqu'il faut. 4 mois plus en mai, il passe, vous savez le PJ le Concorde pays c'est en 2 temps, il passe le premier temps pendant l'école tout le monde le passe, il y a ceux qui l'ont, il y a ceux qui ne l'ont pas. Ce qui ne l'ont pas ils sont gardiens de la paix classique comme aujourd'hui, ceux qui l'ont, ils ne sont pas au PJ, ils peuvent passer juste après la formation initiale qui prévoit déjà un long stage la deuxième partie, et une fois qu'ils l'ont, que dit le texte, c'est grosso modo 30 mois on n'est pas super loin. Des trois ans d'aujourd'hui 30 mois où on les teste, on regarde si effectivement ce sont des bons officiers de police judiciaire, je pourrais dire adjoint ou stagiaire avant d'être définitivement des OPJ, on ne met pas, contrairement à ce que j'ai entendu il a quelques instants, c'est méconnaître le texte que je vous propose, on ne met pas les gens directement sans. Si d'école comme OPJ, on leur fait passer 30 mois 30 mois donc dans quelle activité professionnelle notamment la statut de la fonction publique, on fait passer des gens 30 mois l'expérience de on confirme OPJ et puis à la fin des fins, monsieur Ben arrange ce que vous dites, pardon, est à la fois juste et vous vous dites, ils ont plein de pouvoir bien sûr, mais ils l'ont toujours sous l'autorité du procureur on aurait public, ça se passe tous les jours Monsieur Menage ou le procureur de la République convoque l'OPJ lui dit : vous avez fait de bêtises vous retire votre PJ, ça arrive tous les jours et donc, quoiqu'il arrive, ce n'est jamais un pouvoir absolu donné aux policiers et aux gendarmes, c'est toujours des gens qui justifie des actes qu'ils font et notamment lorsqu'il ne serait pas digne de cet acte lorsque le l'autorité judiciaire du coin n'a plus confiance en lui, on peut retirer cet OPJ sans que la police, gendarmerie, 10 puisse dire quelque chose, moi je vais vous dire il faut être cohérent dans la vie politique, vous pouvez pas à la fois tous constaté qu'il manque des OPJ en France, il en manque à peu près cinq mille tous me dire les violences intra-familiales, ça ne va pas assez vite, on vous n'écoutez pas assez les gens vous faites ne fait pas cette procédure, vous donnez pas ça, ah, c'est à la justice tous m'écrire pour avoir des OPJ dans mon département et puis quand j'arrive avec une solution structurelle qui a été discuté avec tous les syndicats de police, avec l'ensemble de la magistrature par le garde des Sceaux, trouver un compromis qui est présenté devant vous dire : ah ben non

moi je suis désolé je pourrais également lorsque j'ai eu 22 23 ans passé un concours de commissaire de police ou un concours de gardien de la paix, un concours de l'École nationale de magistrature et s'il est choisi, l'École nationale de la magistrature, j'aurais eu 22 23 24 ans, je serai sortie après, comme l'a très bien dit Marc-Philippe Daubresse hier un taux d'école à peu près similaire et j'aurais de substitut du procureur, immédiatement et je crois qu'un substitut du procureur, immédiatement, le procureur de permanence, il a des pouvoirs beaucoup plus important pour la liberté de chacun. Que le simple officier de police judiciaire, excusez-moi, ce constat. Et vous ne faites pas ce procès, personne n'a prévu que dans le code de procédure pénale, les magistrats doivent en 3 ans d'expérience avant d'être substitut non on considère tout ce que les policiers se quand même un peu plus qu'on compte les autres. Quoi, si je vais écouter cette démonstration moi, je me refuse à penser que les policiers sont plus qu'on coupe les autres. Merci, Monsieur le Ministre, je mets donc aux voix, c'est 4 à Monsieur Gaudin Roche pour explication de vote. Je vais pas redescendre sur le fond, ces amendements, je voulais juste dire à Monsieur le Ministre, que plutôt que de faire une loi d'exception qui vous permettrait d'être au pays, je pense que si jamais vous aviez des volontés ou des velléités je pense que vous feriez un très bon conteur d'histoires, parce que vous savez que c'est ce qui ce qui est extraordinaire, je me, je vous le dis, mais vraiment toutes, il y a, il y a aucune velléité de de polémique là-dedans ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que nous développera des arguments et c'est pas le premier amendement sur lequel nous des développant

conclusion de nos arguments pour dire : ben voilà, on n'a jamais dit que les policiers étaient plus qu'on croit que les autres, excusez-moi de vous le dire ça c'est vous qui le dites, c'est pas moi c'est votre expression, par exemple, vous nous dites : on n'a pas dit de politique cohérente monsieur midi Doudou, pensant que nous avons politique aussi cohérente que la vente mais je critique pas la cohérence de la vente de critiquer pas la cohérence de la nôtre, ces 2 exemples que je prends juste la dans la dernière expression que vous avez fait, mais je pourrais en citer pas mal, j'ai pris des petites notes. Merci, je mets donc aux voix ces quatre amendements avec 2 avis défavorables qui vote pour. Qui vote contre. Ils ne sont pas adoptés jamais aux voix, l'article 9 qui vote pour, contre, abstention il était adopté, nous passons à l'article 10 avec de prises de parole Madame Conconne. Madame la présidente, monsieur le Ministre, oui je vous avoue que j'ai été très satisfaite de découvrir dans cette loi Lopmi cette fonction d'assistant, ces personnes qui peuvent être à côté de nos fonctionnaires de police souvent submergé de travail et de travail administratif cependant quand j'ai questionné un certain nombre de professionnels aussi bien au niveau du parquet qu'au niveau de, de la police, j'ai senti quelque réticence qui seraient ces personnes quel est leur niveau de professionnalisation d'expertise, et cetera, la même hein pour la boutade et là, c'est juste pour vous faire sourire, qui m'a dit : j'espère que ce seront pas des petites stagiaires qui vont se charger de la photocopie et du café, donc Monsieur le Ministre, j'aimerais que vous puissiez me rassurer

souvent de fréquenter les commissariats et j'ai pu voir comment les professionnels étaient submergés de travail, des tendances à courir partout, recueillir des preuves, y a des copies téléphoner et cetera si à quelqu'un qui peut les aider en tout cas pour moi ça a été une bonne idée, maintenant, il vous appartient de me rassurer de nous rassurer collectivement sur ce niveau d'expertise et de professionnalisation de ses adjoints assez ces professionnels de police. Si cher collègue Madame Benbassa. Si présidente, monsieur le Ministre, hein, chers collègues, oui, et la procédure pénale est des plus complexes dans notre pays, oui l'accomplissement des tâches qui en découle et fastidieux oui la formalité de certaines d'entre elles peut pousser à l'exaspération, par conséquent, oui la procédure pénale et chronophage pour les officiers de police judiciaire non l'intention des réformes successives ne fut pas de rendent plus dur de leur travail, non la mission de ces officiers ne se cantonne pas à l'exécution de démarche formelle, enfin non, l'investigation ne doit pas souffrir d'un manque de temps pour autant l'efficacité des enquêtes ne peut être mesurée par le seul calcul du nombre d'heures passées sur une opération qu'elle soit liée au fond ou à la forme, c'est pourtant l'intention de cet article, vous proposez monsieur le Ministre de décharger ses officiers de police judiciaire d'une partie de leurs missions au profit d'assistant d'enquête. Or, certaines d'entre elle nécessite une appréciation particulière, c'est le cas par exemple de l'interception des correspondances le réalisation exige, comme le remarque le Conseil d'État que ne soit seulement retranscrit les éléments utiles à la manifestation de la vérité, les officiers de police judiciaire ont alors une fonction importante dans cette procédure, nous ne devrions pas la déléguée à des assistants d'enquête qui n'ont pas la même formation que ces officiels merci beaucoup. Merci, nous passons à l'étude de trois amendements de suppression identiques Monsieur Bénard 59. Merci madame la présidente, ça va pas être très populaire dans plus sa suppression le le le présent amendement a pour objet, effectivement, de supprimer cette nouvelle fonction d'assistant d'enquête de la police judiciaire. Techniquement, cette nouvelle fonction implique le déploiement de personnels formés juridiquement, bon c'est très bien, elle pose quand même des questions sur le rôle de ces agents et sur la nature et l'ampleur du contrôle qui s'exercera sur leur activité, c'est le sujet que nous voulons poser. Je vais citer une seule personne mais je pourrais citer plusieurs c'est c'est le professeur Olivier Kahn, professeur de droit, qui a exprimé ses inquiétudes quant à la création de ses nouvelles fonctions le risque est-ce que ce greffier, entre guillemets, puisque c'est un peu la fonction qu'il y a été défini

quels seront les moyens octroyés aux juridictions à la Défense pour s'assurer que telle n'est pas le cas, qui habilitera les greffiers et à quelle autorité sera-t-il soumis, quelle sera la responsabilité des greffiers, à raison de leur acte la régularité de ses actes de procédure de ses agents interrogent également aussi le Conseil des barreaux, qui crée une forte augmentation de procédure pour nullité des actes d'enquête réalisée par ces nouveaux assistant, ce qui irait donc à l'inverse, a contrario de de l'objectif recherché la création de postes nouveaux de personnes moins rémunérés et qui aura un statut inférieur à celui des agents des forces de l'ordre qui devront fournir un travail tout aussi exigeant que celui mené par les OPJ les APJ ne nous paraît donc pas la solution adéquate pour pallier le manque d'effectifs au sein de la police judiciaire enfin cette nouvelle fonction au statut un peu flou, ne nous semble pas offrir toutes les garanties de conscience d'explication de la procédure qui sommes nécessaire lorsqu'il s'agit de convoquer une personne à un entretien en vue d'une audition, la sous-traitance de mission et d'actes essentiels au bon déroulement de la procédure d'enquête ne nous paraît donc pas acceptable en l'absence de ces précisions et d'expérimentation existantes de ses assistants d'enquête nous demandons donc la suppression de cette mesure. Monsieur Favreau, l'amendement 169. Porte là un nouvel amendement de de suppression, j'ai brassé pas mal de procédure dans ma carrière et je sais à quel point la qualité de l'élaboration de ces documents est essentiel pour la suite des procédures qui vont généralement devant le tribunal je pense que là on est en train de décrédibiliser peut être le le travail de la police, qui à ce jour, a une réputation qui n'est plus à faire et que on va offrir en quelque sorte au juge des procédures qui peuvent éventuellement présenter des carences d'ailleurs, le Conseil d'État a exprimé de vives réserves sur le Champ d'intervention de ses assistants d'enquête dans les avis qui l'a vendu en mars et en septembre 2022, c'est la raison pour laquelle je demande la suppression de cet amendement. Merci madame la présidente Assassi amendement 193. Oui merci madame la présidente, écoutez, on va aller dans dans dans le le le même sens, mais je ne me permettrais à ce stade de, de, d'être la porte-voix en fait du des inquiétudes de porter la voix pardon du CNP et donc d'exprimer du Conseil national des barreaux et et d'exprimer leurs inquiétudes et je le fais d'autant volontiers que je partage leur inquiétude et que distille, ils nous disent que que la notion d'assistant d'enquête et pour eux, en tout cas, c'est ce qu'ils ressentent dans leur profession et est un facteur de dégradation de la qualité de l'enquête par la création donc de cette catégorie d'assistant d'enquêter et il rappelle que l'assistant d'enquête ne peut procurer toutes les garanties d'un OPJ en terme de respect des droits de la défense, de respect de la procédure, ou encore d'explication ou au plaignant au plaignant ou à la victime et que cette nouvelle fonction va créer un corps intermédiaires aura pour effet d'ajouter une énième lourdeurs administratives et il rappelle, comme vient de le faire, notre collègue que le Conseil d'État a fait part de ses réserves dans ses avis de Mars et de septembre 2022 sur le sujet. Monsieur le rapporteur, votre avis. Madame la présidente, sur ces amendements identiques et proposant la suppression de de l'article, je voudrais dire que le Conseil d'État effectivement pointé la nécessité que les transcriptions d'enregistrements reste complètement sous le la responsabilité des officiers de police judiciaire, Didier, agent de police judiciaire pour répondre à cette critique, la commission a adopté un amendement notre collègue Alain Richard, qui propose de mieux encadrer cette procédure et dans le dispositif lui-même et l'étude d'impact, détaille déjà les modalités, nous avons prévu de plus que sera menée dans les 3 ans, une évaluation de cette réforme qui permettra dans la dans mesurer la l'intérêt éventuellement les limites, et par suite d'apporter les correctifs nécessaires dès lors nous, nous ne souhaitons pas la suppression de cet article, notre avis est défavorable. Merci, monsieur le Ministre. le rapport préliminaire de de notre nos articles de loi mais je voudrais redire 3 3 choses rapides. La première, monsieur Favreau c'est que le Conseil d'État, s'il a émis des critiques et des réserves n'a pas souhaité d'joindre le disposition, il a donc considéré conforme à la Constitution à notre état de droit, il a demandé que nous puissions avoir. Des précisions précisions qui seront apportées, puisque tous les décrets qui sont évoqués dans le texte de loi sont des décrets en Conseil d'État, donc je veux dire d'abord au Parlement : premièrement, que tout ce qui concerne concerne les assistants d'enquête parce que ils touchent à la procédure pénale seront vus. essayer de le faux par le Conseil d'État, il n'y a pas de décret simple. Je pense que ça peut rassurer une partie de nos discussions, le 2ème point : il ne s'agit pas, monsieur le sénateur, de pouvoir faire faire n'importe quoi, 6 ans d'enquête et de les laisser ainsi remplacé j'ai bien compris que vous ne n'étiez pas forcément contre la lettre du texte mais contre éventuellement son application qui pourrait amener un certain nombre de personnes à faire des choses différentes de ce que lichette voudrez puisque nous avons listé dans un article assez long malgré tout. Mais c'était nécessaire pour justement vous rassurer, ce qu'il pouvait faire, et d'ailleurs, on peut le lire ensemble

il y a bien sûr procès de transcriptions des enregistrements qui sont prévues dans le code de procédure pénale, il y a de la réquisition des images de caméras de vidéo-protection il y a la convocation de toute personne qui va être entendue par justement un officier de police jeudi. Pierre et l'interprète donc qu'est-ce qui va faire cet assistant d'enquête, il va faire le greffier, comme vous l'avez très bien dit, il va faire la forme de l'enquête, il ne fera pas le fond de l'enquête, encore une fois, je prends parallélisme avec la magistrature, personne ne s'inquiète qu'il y a des greffiers et que ces greffiers appellent l'avocat fasse des photocopies, rappelle un certain nombre de dispositions demande des ampliation, des dossiers, mais c'est pas le greffier qui interroge des personnes, le greffier par nature, il s'occupe de la forme et c'est bien le juge d'instruction qui s'occupe du fond et on sait tous que greffier là une part très importante, il est évidemment conditionné ce greffier par une forme de statut de talent de sa formation et ce que nous devons regarder avec monsieur le rapporteur, qui l'a très bien dit, c'est qu'elle est la formation, quel est le statut de ces personnes madame Assassi, vous devriez être sensible, alors j'entends que nous sommes tous sensibles évidemment au aux remarques du Conseil national des barreaux, je les prends ma avec beaucoup d'intérêt mais vous pourriez aussi être sensible par le début de l'article et c'est là où je vais faire la sénatrice communiste à votre place. Si vous me si vous me le permettez puisque je constate que je suis le seul à m'inquiéter du statut des ouvriers de la sécurité, comme dirait votre candidat à la présidentielle pour qui j'ai de l'estime, je me permets de reprendre l'article. c'est même le début qui devrait vous faire plaisir et je m'étonne que une sénatrice communiste défendent les avocats en dépit des agents de la fonction publique, les assistants d'enquête sont recrutés parmi les militaires du camp de soutien technique administratif de gendarmerie nationale et les personnels administratifs de catégorie B, de la police et de gendarmerie nationale et là c'est pour monsieur Ménard Roche ayant satisfait une formation sanctionnée pour un examen certifiant leur aptitude à assurer l'émission que la loi leur confie. C'est-à-dire que je regarde le le le le l'armée du personnel administratif, technique et scientifique de la maison, police et gendarmerie, je leur dis pendant très longtemps, vous avez été considéré comme la 2ème roue du carrosse des rémunérations en baisse, vous êtes des agents de catégorie B, des difficultés très forte faire entendre de la communauté de la gendarmerie nationale et de la police nationale et jamais on vous met en avant, alors que vous faites tous les jours des choses extrêmement importantes dans un commissariat, une brigade de gendarmerie et je dis je, je, je, je puise chez vous, hommes et femmes de bonne volonté, jamais reconnu par la fonction publique, la capacité de vous élever d'aller vers des fonctions de catégorie A part méritocratie sans jamais aller voir des contractuels ou je ne sais quel autre facéties dont vous pourriez aisément m'accuser dans d'autres circonstances, et je dis avec une formation qui va prendre en charge ou le ministère de l'Intérieur, on va vous faire monter en compétences pour pouvoir accéder à une belle fonction qui, celle de l'assistant d'enquête, donc quelque part, j'ai un peu l'impression, madame la sénatrice de faire ce que vous aviez rêvé. si je peux me permettre, monsieur je je vous permets, madame la présidente, allez-y, non mais c'est pour répondre à Monsieur mini-je je connais son humour maintenant en tout cas je perçois mieux vous comprendrez bien que moi aussi je suis très satisfaite que vous soyez très attentifs au statut de la fonction publique, mais moi je n'oppose pas le statut de la fonction publique et les autres professions de la de la fonction publique, que ce soit le statut de la fonction publique d'État ou de la fonction publique hospitalière, je suis pour la, comment dire, la modernisation et le développement de ses statuts et surtout l'élévation des salaires de ses personnels. Merci, je mets donc aux voix ces trois amendements avec 2 avis défavorables qui vote pour. Qui vote contre. Qui s'abstient, ils ne sont pas adopté 2 amendements qui font l'objet d'une discussion commune Monsieur Durin, le numéro 36. Oui merci madame la présidente, là, moi je n'ai jamais rêvé d'être une sénatrice communiste, en revanche, j'essaie de réfléchir comme peut le faire le le ministre de l'Intérieur qui est assez taquin, cet après-midi, alors comme on arrive pas à faire passer nos amendements de suppression, on s'est dit on va faire autre chose et donc là, on essaye d'aller dans le détail, vous avez dit monsieur le Ministre, que les assistants d'enquête allait avoir une longue liste d'de choses à faire, et d'ailleurs, effectivement dans le texte il y a 8 points qui sont énoncés hé ben on vous propose parce que ça va faire beaucoup de travail dans supprimer, hein, le huitième et ce ce 8ème point que concerne-t-il, concerne la transcription des enregistrements prévus par les articles 100 tiré 5 du code de procédure pénale et 7 senti tirer 95 18 du même code pourquoi nous interrogeons-nous sur ces enregistrements, il est dit que que ne doivent être retranscrit que les éléments utiles à la manifestation de la vérité et on comprend bien que chez c'est presque greffier de police c'est assistant d'enquête vous souhaitez vont dégager les OPJ qui vont dégager du temps de travail pour les OPJ or sur la transcription des éléments que pourrait être amenés à à faire les assistants d'enquête, quelle est la part de ce qui relève de l'enquête, quelle est la part de ce qui relève d'une transcription formelle et est-ce que on peut vraiment distinguer finement entre ce qui est utile à la manifestation de la vérité et ce qui n'est finalement qu'une transcription mécanique d'éléments de contenu, et il nous semble que il serait prudent de ne pas leur confier cette tâche. Merci.

on va essayer d'aller encore un peu moins loin donc d'aller encore un peu plus dans le repli, donc moi j'ai supprimé que 2 des alinéas Jérôme supprimer trois j'en ai supprimé avec deux qui concerne exactement le même poids que Jérôme Durain voilà messieurs qui paraissait dans dans dans le texte, c'est-à-dire les alinéas 36 et 39 ce qui concerne effectivement les procédures de transcriptions des enregistrements prévue par l'article 105 et 706 95 18 du code de procédure pénale là d'ailleurs, le Conseil d'État, il est très critique sur ce point, d'ailleurs, et donc c'est un des points sûrement auquel vous avez fait allusion tout à l'heure en disant que, il y a un certain nombre de, de, de choses qui qui se fait en fonction de cet avis là et donc nous en ce qu'on demande en fait à ce que les transcriptions des enregistrements restent de la compétence des OPJ ou des API tout simplement et je sais pas, j'espère que c'est un un amendement de repli a minima par rapport au à l'autre, a une petite chance peut-être d'avoir un avis favorable. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces deux amendements identiques, mais pas. Madame la pas tout à fait identique le Conseil d'État effectivement pointé la nécessité que les retransmis, création de 2 enregistrements reste sous la responsabilité des OPJ ou des ou des agents de police judiciaire, la commission a adopté, je le disais tout à l'heure, un amendement à l'initiative de notre collègue Alain Richard pour mieux encadrer ce dispositif ce ce point dont le dispositif lui-même et l'étude d'impact tailles déjà les les modalités. Dès lors, il nous semble que le risque pointé par le Conseil d'État semble écartée et sous l'autorité des OPJ, ça veut dire que l'officier de police judiciaire va indiquer précisément ce qui notamment le audition est intéressant et mérite d'être retranscrit. Donc je pense que les garanties sont suffisantes dans dans la rédaction qui est proposé par la commission des lois. Merci, Monsieur le Ministre votre même avis. alors qu'on sait tous que lorsque vous faites une audition à l'exception, j'ai dit pour les auditions, qui concerne les mineurs dans les violences sexuelles sont toujours des synthèses des réponses, je sais pas si vous avez eu le le le le l'occasion d'être auditionné par un service de police ce n'est jamais l'intégralité des propos que vous tenez qui sont retenus, y compris par l'officier de police judiciaire qui est en face de vous, et d'ailleurs, c'est tellement vrai que on fait relire. Ah vous même la personne qui était auditionné à votre avocat si vous accompagne et puis de c'est l'OPJ lui-même qui signe des questions et les réponses et vous avez le droit de changer telle ou telle terme évidemment tant que personne n'a signé l'audition le il a déjà quelque chose qui relève de la synthèse, c'est pas un PV de synthèse mais ça relève de la synthèse en l'audition d'abord je voudrais vous rassurer, chacune et chacun, ça n'a pas été dit mais peut être que ainsi votre amendement serait superfétatoire, c'est bien l'OPJ qui signe. C'est pas la PJ qu'ici, donc là, BJ, vous comprenez bien qu'il ne fait pas l'audition, c'est pas lui qui pose des questions et il ne signe pas, il est l'assistant de l'enquêteur, comme son nom l'indique, mais comme le juge d'instruction et celui qui pose des questions, alors là, le juge d'instruction même, contrairement à son enquête, puisque c'est les greffiers, greffiers, ils ont des ordinateurs et il voit en Direct ce qui se fait sur ces ordinateurs et à la fin, c'est bien le juge qui signe et pas le greffier enfin le greffier peut signer puisque c'est un formalisme encore différent de la police nationale et gendarmerie nationale au Gabon, je vous rassure, hein, ça existe déjà de l'OPJ si troisièmement, vous l'avez vous-même entendu je crois dans le Beauvau de la sécurité qu'est-ce qu'on essaye de faire part ça demain, mais dans les et messieurs les sénateurs, il y aura, et c'est heureux, des retranscriptions il y aura des propos que nous tiendrons parce que les assistants vocaux vont permettre de faire gagner beaucoup de temps à chacune et à chacun, le policier posera la question, la personne répondra et comme votre logiciel Siri sur votre iPhone mais ce sera beaucoup plus efficace, puis c'est déjà vrai dans beaucoup de chant, de la vie économique et administrative, il y aura une retranscription on gagnera ainsi énormément de temps, il faudra corriger un certain nombre de fautes de syntaxe, par exemple, mais aussi et c'est l'objet de notre discussion d'aujourd'hui ben formaliser à un certain nombre de sujets pour qu'il soit en lien avec l'interrogatoire qui vient d'être menée, donc ce que fera demain l'assistant d'enquête on ne va pas changer de loi tous les jours, c'est de regarder comment fonctionne cet ordinateur de retranscription de corriger les les fautes de ponctuation, les fautes d'orthographe qui pourrait avoir lieu de synthétiser à Saint-nombre de choses et de soumettre à son OPJ qui lui seul va relire et signer la procédure ce sujet donc vraiment, je voudrais vous rassurer, si c'était les explications que vous étiez à voir, il ne s'agit pas de remplacer le PJ par cet assistant d'enquête qui pourrait lui-même retranscrire puis signer sans jamais qu'enquêteur. En 2 la procédure, il s'agit d'un assistant d'enquête qui ne fait qu'assister sans jamais être le responsable n'y a ni de Z de la procédure. Merci monsieur le ministre monsieur Richard pour explication de vote. C'est le président, Monsieur le Président, je voudrais compléter le le débat en insistant sur le sujet de la retranscription des écoutes, je n'ai jamais vu personnellement le texte, je n'écoute ni d'ailleurs entendu le son, mais j'ai rencontré un certain nombre de gens qui m'en parlé la retranscription d'une écoute est un travail assez fins parce que évidemment les gens qui se parlent dont on recueille le son dans un autre contexte, s'exprime suivant les habitudes de langage qui sont pas forcément celle de la procédure pénale, employes de Largo bascule de temps en temps, dans un langage étranger il y a des silences et cetera, donc le travail d'interprétation est important votre amendement m'amène à apporter un tout, une toute petite Pierre aux travaux préparatoires ni à la préparation du décret du Conseil d'État, il est évident que dans la conception de l'encadrement

il ne peut faire que du brut en quelque sorte dire recopier l'ensemble des des mots les son employé, et ce sera bien l'officier de police judiciaire, parce que ça c'est de la vraie matière pénale pénale il des facteurs qui sont incriminant ça ne peut être que l'officier de police police judiciaire qui fait une synthèse, une remise en français qui aura le caractère d'un document probant.

Très bien, un amendement de coordination, monsieur le Ministre favorable je mets donc aux voix cet amendement avec un avis favorable du gouvernement qui vote pour. Contre, abstention il est adopté, je fais voter donc l'article 10 ainsi modifié qui votent pour, contre, abstention il être adopté je mets aux voix, l'article 10 bis qui vote pour, contre, abstention-il être adopté, nous passons à l'article 11 avec un amendement numéro 194 présenté par la présidente.

gêne beaucoup c'est qu'il prévoit de modifier l'article 60 du code de procédure pénale, en prévoyant que les OPJ puisse procéder à des constatations et des examens techniques ou scientifiques sans qu'il soit nécessaire d'établir une réquisition à cette fin, ce qui pendant l'enquête, éloigne les enquêteurs du contrôle du contrôle en temps réel du parquet ou du juge d'instruction, il est difficile donc d'accepter l'idée que la police technique et scientifique puisse s'auto-saisir la de la disposition et donc flou et ne précise pas l'encadrement primordial de la procédure de réquisition pour les nécessités de l'enquête, la validité de la procédure risque donc de se retrouver atteinte. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis. Monsieur le rapporteur. dans le cas des enquêtes préliminaires ou de ou de flagrance l'obligation actuelle faite au service en charge de l'enquête de procéder à une réquisition judiciaire pour solliciter les agents de police technique et scientifique, afin qu'ils effectuent des investigations techniques et scientifiques ou une copie de l'informatique sur un support placés sous scellés, nous avons décidé en commission de compléter tandis en clarifiant les procédures de recours à la police technique et scientifique, en particulier s'agissant des analyses réalisées à l'issue de prélèvements génétiques ou papi air il s'agit d'un article très attendu par les services de la police scientifique et technique, qui va dans le bon sens, celui d'une meilleure efficacité sans affaiblir les garanties offertes aux droits et aux libertés, notre avis défavorable à la suppression de cet article. Merci, monsieur le Ministre, même avis. Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Contre, abstention, il n'est pas adopté, monsieur le rapporteur, l'amendement 229 au nom de la commission des lois. Il est de coordination, madame la présidente. Très bien, Monsieur le Ministre votre avis favorable je mets donc aux voix cet amendement avec un avis favorable du gouvernement qui votent pour, contre, abstention il est adopté. Je fais donc voter sur l'article 11 ainsi modifié qui vote pour. Contre, abstention-il être adopté, nous passons à l'article 12 avec l'amendement 195 présenté par la présidente. Oui merci madame la présidente, cet amendement donc vise à supprimer la création d'une présomption d'habilitation à la consultation des fichiers de police institué par l'article 12 du projet de loi au motif de simplification nous considérons ici qu'il est dangereux de concevoir que la loi puisse créer une cause d'exonération de nullité même issu d'une absence de mention d'habilitation qui est pourtant une garantie de fiabilité d'une procédure, on ne peut admettre l'idée qu'un agent non habilités puissent agir sans que cette action ne puisse ne puisse impacter la validité de la procédure, cette brèche juridique dans les règles applicables en matière de nullité, avec ou sans texte cause une atteinte excessive aux principes fondamentaux, la loi actuelle qui prévoit une cause de nullité s'il existe un grief suffit, selon nous, à répondre aux objectifs de sécurité juridique poursuivi. Si madame la présidente, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Oui. Oui, madame la présidente, madame la présidente, si vous savez que la question des fichiers relève chez moi parfois du trouble obsessionnel compulsif, mais néanmoins, je trouve que faute avouée à moitié pardonnée, mais en tout cas c'est vrai que je suis très sensible à cette question là pour autant ne cette simplification est la bienvenue et la maman vous proposer un amendement de suppression, en réalité, il s'agit d'alléger des obligations formaliste qui n'apporte pas de véritables garanties en soi, le juge ayant toujours la possibilité de vérifier la réalité l'habilitation et j'ai j'ai je crois pouvoir dire sans me tromper que parfois, c'est le fait de ne pas préciser cette habilitation peut faire capoter la procédure donc c'est il y a, il y a un élément formelle, c'est hyper formel sa raison pour laquelle, bien qu'ayant ce trouble sexuel compulsif, j'ai pensé que c'était une bonne chose de maintenir cet article dans le texte. Merci monsieur le ministre. je, je veux dire un mot, madame la présidente, parce que je, je comprends très bien la question autour de la consultation des fichiers qui est une un encadrement bienvenue de la part du du parlement et sans ce que le rapporteur Hervé par ailleurs membre de la CNIL lorsqu'il donne un avis favorable devrait vous rassurer, je sais pas, cependant vous dire pourquoi on fait ça, la consultation des fichiers pour le ministère de l'Intérieur, passe par une plateforme qui s'appelle Cheops qui elle-même sécurisé, les agents du ministère Intérieur ne ne peuvent pas aller sur cette plateforme donc ils n'ont pas rentré leurs badges et leur numéro qui identifie la personne et donc si je veux dire, il ne peut pas y avoir de personne sauf à trahir profondément le droit et à seront évidemment responsable d'un délit très grave qui est évidemment poursuivi, il peut pas y avoir de personnes qui ne soit pas habilité qui consulte ces fichiers. Pour autant, nous constatons beaucoup de nullité dans des procédures de personnes qui n'ont pas formé, l'habilitation formelle, alors qu'elle est de droit. Donc ce serait un peu, c'est un peu dommage de faire tomber des procédures où on doit mettre en prison des criminels pour de de simple nudité, que les avocats extrêmement compétent, remarque évidemment, mais qui ne touche à rien, à la protection des individus donc objectivement, madame la présidente, je crois que toutes les garanties de consultation des fichiers sont sont portés et simplement c'est plutôt une garantie qu'une procédure aille jusqu'à son terme. C'était favorablement. Vous êtes donc défavorable, monsieur le Ministre. Je mets donc aux voix cet amendement avec un TOC favorable Star du rapporteur et un avis défavorable de la part du ministre qui vote pour. Qui vote contre. Qui s'abstient, il n'est pas adopté 2 amendements identiques monsieur Durin l'amendement numéro 37, monsieur le président, Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai bien attendu les explications de monsieur le rapporteur et de Monsieur le Ministre, notre amendement se borne à la suppression d'une phrase, mais elle est importante et monsieur le Ministre, vous nous dites que ça va simplifier les choses, je veux bien le croire toutefois la création d'une présomption d'habilitation au motif de la simplification procédurale contourne de manière explicite le principe selon lequel l'habilitation des agents accéder aux fichiers de police constitue une garantie pour la protection des libertés individuelles et même et ne peut donc pas être présumé, je vois bien l'intérêt des badges de toute nature, d'ailleurs, tout le monde et badgé constamment à tout propos et quelques fois hors de propos, là il s'agit de procédures judiciaires pour lesquels des garanties sont. Demandez sont exigés et je crois qu'il convient de rester extrêmement vigilants sur ces questions, la règle, fondée sur le contrôle de l'habilitation constitue en effet avec celles relatives à l'authentification et à la traçabilité, un élément essentiel de la sécurité des données personnelles, elle permet d'écarter toutes les consultations régulières, c'est là que la raison pour laquelle l'acte d'un agent qui consulte un fichier de police sans y avoir été expressément habilitée conformément aux prescriptions de l'acte réglementaire autorisant la création de ce fichier entache la procédure d'une nullité d'ordre public et si Monsieur le Ministre, vous avez raison de dire qu'il y a des avocats intelligent et vigilants et sourcilleux, je sais qu'il y a aussi un grand nombre de policiers intelligents vigilants et sourcilleux. Merci monsieur. Ben, amendement 67. écoutez, c'est, c'est la même, la même raison, le même amendement effectivement que que celui qui vient d'être défendu, donc je je rajouterais juste qu'effectivement nous trouvons qu'un certain nombre de formalisme sont pas superflu, qu'il s'agit souvent de garantie de de droit et que donc voir une simplification juste sous la sous le prisme uniquement d'une accélération n'est pas forcément bénéfique, donc nous soutiendrons effectivement cet amendement, qui est le même que celui que vient de soutenir monsieur Merci, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Oui, madame la une présidente même démonstration que pour l'amendement, qui que vous avez soumis au vote : avis défavorable. Monsieur le Ministre, ma ma vie. Merci, l'avis du Conseil d'État qui a été cité précédemment, qui a même dit joint le l'article AFD dont on parlera après, n'a pas eu à à redire sur la suppression de habilitation, ce qui devrait quand même nous inspirer toutes et tous soit dispense accordée aux forces de l'ordre, le projet de loi insère dans le code de procédure pénale Arctique, hein, 5 nouveaux qui dit ne pas rappelle que seuls les personnels spécialement, individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitement au cours d'une enquête ou d'une instruction et dispose que la réalité de ces habilite de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlé à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande, en particulier de la mention de cette habitation ce différentes pièces de procédure résultant de la consultation, ce traitement ne saurait emporté par elles-mêmes nullité de la procédure, les mêmes règles sont introduits dans le code des douanes d'obliger de la mesure et de dispenser les agents de l'obligation de produire, elle est conforme à nos jurisprudence de la Cour de cassation, elle cite notamment le Conseil cite la chambre criminelle du 19 février 2019 donc. Une jurisprudence assez récente, et le Conseil précise que l'accès des données personnelles contenues dans ces fichiers aux seules personnes régulièrement autorisée et au nombre des garanties exigées par la directive de l'Union européenne, je vais terminer, madame la présidente à l'égard de vêtements données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention, une section d'infractions pénales d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales à la libre-circulation permet d'être vu par le présente articles déposés par le projet de loi et donc le Conseil conclut. Si l'absence de l'habilitation versé au dossier ne pourra plus en vertu du projet, être à elle seule une cause de unité de la procédure, l'absence d'habilitation d'agent ayant consulté les données, comme le rappelle le projet demeure quant à elle, puisqu'il s'agit pas de supprimer toutes les habilitations quant à une cause de nullité qu'il appartient à personne concernée, le cas échéant aux juridictions compétentes de soulever dans des conditions prévues par le code de procédure pénale, donc ce qu'on supprime, c'est bien l'habilitation générale mais bien évidemment la question d'invitation particulière et toujours une cause de nudité, c'est sans doute pour cela que le Conseil d'État et moins sourcilleux que vous, monsieur le Président sur.

Qui vote contre. Qui s'abstient, ils ne sont pas adoptés j'ai mets aux voix, l'article 12 qui vote pour, contre, abstention il est adopté, nous passons à l'article 13 avec 2 amendements identiques de suppression monsieur Bena Roche le 66. les instructions générales permettent de requérir des données sans contrôle préalable d'aucune entité, que ce soit même du procureur de la République, alors les auteurs du présent amendement estime que de telles autorisations générales pose problème à plusieurs égards, d'abord au regard de l'absence de contrôle préalable de ses réquisitions, le droit de l'Union européenne existe déjà, en ce qui concerne les réquisitions de données de connexion à contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante, bien que l'article en cause ne concernent que des données de contenus, celle-ci demeure attentatoire à la vie privée exige a minima le contrôle systématique du procureur de la République ou, au mieux, le contrôle d'une juridiction d'une entité administrative indépendante, tels que les JLD, là encore, une simplification vu comme j'ai dit tout à l'heure sur le seul prisme d'une accélération n'est pas forcément bénéfique ensuite au regard du caractère encore trop générale des données visées par l'article en question qui ne distingue pas suffisamment les infractions en fonction de leur gravité, les données en effet par cette tactique pourra être qui, sur le fondement d'une instruction du parquet dès lors que l'infraction est punie d'une peine de prison ce seuil à parer un peu flou ou peu exigeant en fait les autorisations générales de réquisition des données relatives à lecture à la lecture automatisée des plaques d'immatriculation apparaissent particulièrement attentatoire à la vie privée, car elles permettent la localisation d'une personne au même titre que les données de connexion au demeurant, il apparaît aux auteurs de cet amendement qu'une telle mesure relative aux réquisitions de données ne devrait pas apparaître dans une loi de programmation mais qu'elle devrait être inscrit dans une réforme plus générale des réquisitions de données qui devrait intervenir au plus vite au regard de la décision de la Cour de cassation du 12 juillet dernier. Merci madame la présidente à de nouvelles catégories d'acc. Donc tout ceci a été précédemment argumenter, donc je considère que mon amendement est défendu. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis. Ce sont, madame la présidente des amendements qui visent à la suppression de l'article, les auditions que nous avons menées ont souligné que la mesure était attendue par les acteurs, les différents services de police, de gendarmerie, les magistrats considèrent en effet que l'extension proposée supprime des demandes qui sont chronophages, parfois même déjà utilisée en pratique et permet une simplification la procédure pénale, qui était un objectif de ce texte de loi afin de préserver le pouvoir de contrôle du magistrat parquetier sur les enquêtes, le texte a été modifiée depuis que cette mesure a été proposé dans le projet de loi relatif au parquet européen la justice pénale spécialisée les actes pour lesquels les réquisitions général sont autorisés sont désormais limitativement énumérées par le texte et le procureur de la République sera informé de l'ensemble de des réquisitions afin de pouvoir exercer effectivement son pouvoir de contrôle de police judiciaire, l'avis est donc défavorable. Merci, je mets donc aux voix ces deux amendements avec 2 avis défavorables qui vote pour. Contre, abstention, ils ne sont pas adoptés Monsieur Durand votre amendement numéro 38. Oui, madame la présidente, nous demandons une évaluation nous interrogeons sur le l'intérêt pratique et le gain de temps réel apporté par la possibilité de délivrance d'autorisation générale de réquisition, a priori, dès lors que le parquet doit être informé sans délai au cas par cas de la délivrance de ces réquisitions et être mis en mesure de les contrôler, donc on propose que dans les 18 mois qui suivent l'application de la loi, on puisse avoir un retour sur sa disposition. Alors c'est une une demande de rapport d'évaluation. On voit que le mot évaluation apparaît désormais et c'est c'est stratégique faisait bien considérant la portée réduite de cet article, regarde la pratique existante et de l'extension qu'il opère nous il nous semble peu peu opportun d'envisager un rapport d'évaluation sur un objet aussi restreint. Au surplus, les auditions menées par par vos rapporteurs ont montré que l'article recueille l'assentiment général des différents services de police, les gendarmeries, les magistrats qui, de concert. Considère que cette mesure supprime des demandes chronophage qui pèsent inutilement sur le temps d'investigation et que les autorisations générales déjà existantes permettent une simplification de la procédure pénale est un gain de temps significatif j'ajoute par ailleurs que nous avons parfaitement les moyens de procéder nous-mêmes à cette évaluation en organisant les auditions et où on demandant les chiffres au Ministre qui ne leur ne manquera pas de nous les communiquer avis défavorable. qui votent contre, qui s'abstient il être adopté, nous passons à l'article 13 bis avec 2 amendements identiques de suppression, Monsieur Durand, le quarante-quatre. Alors nous nous intéressons à cet articles bis qui vise à éteindre les prérogatives des agents de police judiciaire, c'est un article qui a été insérée dans le projet de loi à l'initiative des rapporteurs de la commission des lois et il s'inscrit finalement dans une démarche continue d'extension des des attributions des APJ adoptée depuis plusieurs années, démarche qui vise 2 objectifs essentiellement la revalorisation du travail des agents de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire d'une part, et puis d'autre part, la simplification de la conduite des enquêtes en permettant aux et PJ de s'appuyer davantage sur les agents, ce qui devrait être facteur de fluidité dans la réalisation des investigations alors continuer à étendre les pouvoirs enquête des APJ, dans le sens souhaité par cet article, en leur permettant d'effectuer davantage de réquisition davantage d'actes matériels de constatations et notifications sans procéder à une nette amélioration de leurs conditions de formation de bon niveau préalables nous pose difficulté et et nous nous interrogeons sur les garanties qui nous sont apportées en la matière, donc dans le droit fil des dispositions que nous avons exprimé sur les questions d'investigation nous souhaitons par cet amendement, interrogé au fond cette disposition. Si Monsieur le Sénateur Monsieur Bénard votre amendement 65. C'est la même chose, donc je dirais pour résumer ce que vient de dire monsieur durera moins d'expérience, mois de formation, donc effectivement, nous ne souhaitons pas que les rôles soient

En voulant supprimer cet article Madame présidente messieurs du hein et hé ben à Roche s'oppose à l'extension des prérogatives des agents de police judiciaire, que nous avons nous-même introduit en commission, nous avons prévu que l'ensemble des actes réalisés par les APJ seront réalisés sous le contrôle des officiers de police judiciaire en augmentant leurs prérogatives, nous permettons d'organisation des investigations plus souples et à nos yeux. Plus efficace, vous comprendrez que notre avis soit naturellement défavorable. Monsieur le Ministre, même avis je mets donc aux voix ces deux amendements avec 2 avis défavorables qui vote pour. Contre, abstention, ils ne sont pas Z opter amendement 230 monsieur Raoult, coordination, madame la présidente, très bien, je mets donc aux voix cet amendement avec un avis favorable du gouvernement qui votent pour, contre, abstention il est adopté, je mets aux voix, l'article 13 bis hein ainsi modifié qui votent pour, contre, abstention il était adopté article additionnel avant l'article 14 l'amendement 135 et présenté. Il parle Madame Billon vise à améliorer la prise en charge des victimes en posant un délai maximal de six semaines entre le dépôt de plainte et les suites données par le parquet, qu'il s'agisse d'un renvoi devant le tribunal correctionnel d'une mesure alternative aux poursuites ou d'un classement sans suite, trop souvent, les victimes sont confrontés à une attente de plusieurs mois qui les place dans une situation de danger maximal les violences d'un mari ou d'un concubin violent apparaissent ou réapparaissent avec après le dépôt de plainte de la victime, telle est l'objet de cet amendement. La présidente, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Madame la présidente, monsieur le Ministre, l'amendement que la présidente Annick Billon vient de près de présenté est un amendement intéressant en tout cas qui m'interpelle le rapporteur, comme je suis, comme d'ailleurs les amendements Rossignol ou ou tout à l'heure de notre collègue Bazin, ça, ça pose des questions, ceci dit, je suis pas sûr que la réponse apportée par l'amendement soit opportune et d'autre part, comme tout à l'heure, amendement qui qui arrive à un moment donné de la discussion parlementaire où nous n'avons absolument pas la capacité d'en évaluer la portée ni d'entendre les personnes qui seraient concernées par cette par, par cet amendement, je pense en particulier et, naturellement, au 1er chef les au procureur de la République qui seraient amenés à avoir des obligations en termes de délai qui leur ce qui leur seraient imposés, l'amendement pose une vraie question, c'est la question de la motivation des décisions et de la rapidité d'justice dans notre pays cette dommage que nous n'ayons pas pu à l'échelle de ce texte là, interrogé les procureurs de la République, je me demande si c'est tout à fait d'ailleurs le bon véhicule législatif pour parler de ça, je pense que ça coûte encore une fois, ça pourra faire l'objet de discussions dans dans les rapports parlementaires qui sont actuellement

C'est-à-dire que si un hein Madame Kakar avait proposé 15 jours en commission, là, elle propose 6 semaines est-ce que c'est tenable dans le dans les parquets de d'imposer ce type de de délai là et vous observerez qu'il n'y a pas de dispositif coercitif, ça veut dire que si le délai n'est pas tenu. Bah, en fait, le le le le délai il est théorique, on impose un délai au parquet, mais c'est ma foi, si le procureur ne le tient pas ben

elle. Vous êtes du même avis, monsieur le le ministre, très bien parfait, donc je vais mettre cet amendement avec ah pardon, vous avez une explication de vote. il y a cette mission et j'ai à côté de moi une sénatrice en mission désormais pour cette juridiction spécialisée, donc bien entendu on va on on va étudier toutes ces questions, grâce à la mission et Dominique veut rien et sa collègue député donc l'amendement est retiré, je vous remercie. Merci, nous passons donc à l'article 14 avec quatre amendements identiques de suppression monsieur dur hein, vous ouvrez le bal avec l'amendement trente-neuf. Je prends la tête de ce quatuor en faveur de la suppression de cet article, c'est un sujet important que celui des des amendes forfaitaires délictuelles leur généralisation coup elle pose des questions de principe et pour connaître, comme d'autres le retour des acteurs de terrain, il n'est pas contestable qu'un certain on ne de de policiers disent qu'elles leur rendent bien des services en même temps on ne peut pas ignorer le fait que les taux de recouvrement sont pas toujours extraordinairement probant et par ailleurs, les questions de principe qui sont posés et qui valent un certain nombre de de d'organismes ou d'institutions sérieuses comme la Cncdh des critiques sur le dispositif, c'est le le principe d'égalité devant la justice, c'est le fait que cet outil prive le justiciable de garantie assez fondamental le respect du contradictoire, l'individualisation de la peine pour tenir compte compte de la personnalité de l'auteur de l'infraction, sa situation sociale, économique, le recours éventuel à des mesures alternatives par le procureur de la République et sur un certain nombre de sujets, il expose les les justiciables un réel risque d'arbitraire alors. Il faut apprécier le travail qui a été conduit par les rapporteurs qui ont restreint le Champ initial proposé par le gouvernement, on a eu un amendement hier en en commission qui où le gouvernement nous proposer une série complémentaire de délits pour lesquels l'voilà c'est un amendement d'appel au fond sur les principes et qui correspond à un certain nombre de d'interrogations, d'acteurs du terrain qui nous ont vertement sollicité et inciter à ne pas aller dans cette voie.

pour certaines infractions qui ont été listés grâce au travail de notre commission qui dont le rapporteur s'est opposé à la généralisation de l'AFD, il n'empêche que même limité à une énumération de certaines infractions cette généralisation de l'AFD nous pose certains que d'abord, elle relève d'une justice qui nous paraît de moins en moins individualisé ensuite le Conseil d'État, on l'a dit dans son avis du 10 mars 2022 regrettent l'absence de toute évaluation préalable à la mise en place de la FED en France, c'est un sujet si important pour pourtant nous semble-t-il, et je comprends que le gouvernement va y aller vite, mais là le le pragmatisme ou la rapidité ne peuvent pas servir de justification à l'absence d'évaluation des politiques publiques, avant de les généraliser cette absence-là devient en fait de plus en plus fréquentes sur ce texte de loi avant comme sur d'autres et elle devient de plus en plus gênante, s'agissant par exemple des contentieux relatives à l'usage des stupéfiants j'ai j'ai mise nous a donné quelques chiffres, cela étant dit, la réalité c'est que l'objectif aussi consiste. Ah, consisterait à voir s'il y a un effet sur la prévention santé publique est ce qu'il a un effet sur la pratique des consommateurs, donc si il y a un effet sur la prévention, santé publique et la pratique des consommateurs, il y aura forcément un effet aussi sur le trafic, ce n'est pas le cas il y a aucune étude qui le montrent, au contraire, au ils sortent que ça n'en est pas donc, si vous voulez cette évaluation, ce manque d'évaluation nous paraît toujours très compliqué, je rajouterai que, dans ce cas très particulier, il y a quand même un risque d'arbitraire et d'inégalités, les agents verbalisateurs de grands salle s'assurer que les conditions pour verbaliser au moment où il verbalise et apprécier l'opportunité de verbaliser ce qui fait qu'il y a quand même un risque de discrimination de rupture de principe d'égalité devant la justice de rupture d'équité entre les justifiables dans la constatation et la poursuite des infractions pénales, il ne faut pas oublier, c'est le dernier mot, que c'est au procureur l'opportunité des poursuites en matière pénale, selon les dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, c'est pour ça que nous demandons la suppression de 7. Merci monsieur Favreau amendements identiques, ce 170. La présidente, monsieur le ministre, chers collègues, je crois que je je fais miennes les, les différentes argumentation qui viennent d'être développés pour demander l'annulation de cet article, je crois qu'il existe sur cet article un vice majeur, il suffit de regarder la désignation même qui est fait de l'amende forfaitaire, on parle d'une amende forfaitaire délictuelle, qu'est ce qui distingue la contravention du délit en droit pénal, c'est l'élément intentionnel, c'est-à-dire que la contravention, vous n'avez pas à prouver l'élément intentionnel pour pouvoir condamner En matière délictuelle, c'est le cas, et là. Si on relit toutes les infractions qui sont visés, sur cet article, je vois mal comment, à chaque fois que l'élément intentionnel de sera pas prouvé et ce sera pratiquement le cas compte tenu de la façon dont les choses seront présentés, je ne vois pas comment on pourra condamner donc pour cette raison, surtout pour cette raison, je considère que cet article ne doit pas prospérer. Merci madame la présidente, assassine l'amendement 197. Oui merci madame la présidente, donc il notre amendement vise à s'opposer à la généralisation de l'amende forfaitaire des délictuelle pour l'ensemble des délices impuni d'une simple peine d'amende ou d'un an d'emprisonnement, nous souhaitons ici souligné que dans son ah en date du 10 mars dernier, le Conseil d'État s'étaient opposés à la généralisation de l'amende forfaitaire au nom de l'égalité devant la justice, en effet, le Conseil d'État a mis en exergue que le choix de recourir ou non à l'amende forfaitaire reposera sur l'appréciation des agents Werber verbalisateur, il en résultera donc inévitablement en l'absence d'un encadrement un risque d'arbitraire et des disparités de traitement, contraire au principe d'égalité devant la justice pour autant le gouvernement n'a pas supprimé cette disposition, et cette procédure d'amende forfaitaire délictuelle ouvre, selon nous, un risque de discrimination en effet, la Cncdh a récemment souligné que l'amende forfaitaire prive les justiciables de garanties fondamentales coffre la procédure judiciaire en déléguant aux agents de police, une fonction qui relèvent en principe de l'autorité judiciaire, le justiciable ne des de bénéficient dès leur plus de garanties fondamentales telles que le respect du contradictoire, l'individualisation de la peine pour tenir compte de la personnalité de l'auteur de l'infraction de sa situation sociale et économique, ou encore le recours à des mesures alternatives par le procureur de la République ainsi l'amende forfaitaire fait fi du principe d'opportunité de la peine, il s'agit d'une procédure de masse systématiser qui ne fonctionnent déjà pas en terme de régularisation des délits. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. que avec ce projet de loi nous nous risquerions de généraliser les amendes forfaitaires délictuelles, ça me paraît pas être la réalité, nous en avons actuellement droit positif, une dizaine, on y reviendra notamment avec un amendement porté par Sylvia Noël tout à l'heure avec des amendes fait taire délictuels qui fonctionne très bien et d'autres qui posent de vraies difficultés opérationnelles, donc une dizaine dans le droit positif cette dans le texte de la commission et le gouvernement va nous en proposer cette nouvelle, on va passer de 10 à 24. 10 à 24. J'appelle pas sa généralisation parce que si nous avions été dans une logique de généralisation, alors nous aurions pu prendre les 3400 infractions pouvant donner lieu à une condamnation d'un an de prison ferme et là nous aurions été dans une logique totalement différente et nous aurions je pense du côté du du point de vue du Parlement perdu la capacité de décider infraction par infraction, celle qui mérite d'être de donner lieu à la possibilité d'une amende forfaitaire délictuelle, je rappelle qu'évidemment. Ces amendes forfaitaires délictuelles, elle reste sous le contrôle du des parquets et et les droits des personnes mises en cause est totalement garantie, on pourrait revenir d'ailleurs sur un certain nombre d'exemples si vous le souhaitez, mais ça nous a ça à Marc-Philippe Daubresse et à moi-même, au sein des travaux que nous avons mené à la commission des lois, comme quelque chose de proportionner d'ailleurs, on pourra dans l'avenir, en fonction des expériences de terrain retirer des amendes forfaitaires délictuelles ou ajouter de nouvelles amendes forfaitaires délictuelles honnêtement c'est la la l'amende forfaitaire délictuelle qui fonctionne le mieux, qui est celle de, qui est lié aux stupéfiants, c'est 260000 par an, elle fonctionne plutôt bien et heureusement que nos tribunaux ne sont pas engorgé, avec ces amendes forfaitaires délictuelles là et et et ça soulage vraiment et concrètement la justice dans notre pays donc l'avis est défavorable sur l'ensemble de ces amendements de suppression de l'article 14. merci madame la présidente, bon ceci à un moment important de de ce projet de loi puisque il vient compléter la partie simplification de procédure pénale, qui, vous l'avez vu, très fort dans le projet de loi retire le rapport annexé l'essentiel des articles après cyber concerne l'investigation, on l'a vu sur d'enquête, on l'a vu sur les OPJ, nous voilà sur un cadre de simplification pénale que sont les amendes forfaitaires délictuelles, j'avoue, sans faire de politique politicienne, avoir du mal à comprendre la philosophie sur est-ce que les AFD c'est bien, c'est pas bien, puisqu'ils ont été inventés dans par d'autres gouvernements, suivez mon regard, donc je suis pas sûr que ce soit vérité ici est désormais désaccord là, regardons ce qui est pratique et ce qu'il est pragmatique des amendes forfaitaires desquels vous en avez fait depuis longtemps en sécurité routière. Des amendes forfaitaires délictuelles, vous en avez depuis peu de temps, quelques années sur un certain nombre de délits assez simple type la consommation de stupéfiants sur la voie publique, je rappelle qu'il y a des conditions je allais dire monsieur Favreau qui sont à mon avis tout à fait rassurante pour lui d'abord, il faut être avant que 18 ans on met pas de AFD un mineur, il faut être français, il faut ne pas être récidiviste. Il faut avoir une circulaire pénale qui parquet par parquet explique comment l'appliquer, il faut reconnaître le Daily pardon de dire il y a ainsi donc un contradictoire Madame Assassi, c'est pour ça que le Conseil des telle conséquence le le valide et ce sont évidemment des délits que nous vous proposons qui sont objectivement le sang. Acte d'enquête et là où j'ai pas compris votre démonstration, monsieur le sénateur, c'est vous dites une différence entre les contraventions et le délit, c'est qu'il y en a un qui doit être si j'ose dire, encadré dans, dans, dans, dans une enquête et on doit reconnaître l'infraction, c'est le cas de toutes les AFD dont nous discutons aujourd'hui, on peut discuter de la liste, mais pourquoi faire un amendement de suppression dans ces cas-là discutons de l'AFD que vous considérez comme n'étant pas rentrer dans cette case qui consiste, hein, de reconnaître l'infraction de que ce soit un délit objectif je prends des, des, des, des choses par exemple très clair. L'intrusion non autorisée dans une école, bon il y a pas besoin d'actes d'enquête particulier le délit en matière de chiens d'attaque, ceux qui ont été élu local le savent, c'est un un phénomène très complexe et c'est très long, de pouvoir faire condamner quelqu'un qui aurait un chien d'attaque qui n'aurait pas été et et vous évoquez ailleurs que devant les tribunaux, atteinte à la circulation des trains, je dis pour tous ceux qui, notamment en région Île-de-France ou en région lyonnaise sont parfois en attente très longtemps de mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'on avance pas plus vite parce que, évidemment, c'est très complexe, c'est assez facile à avoir une atteinte à la circulation des trains. filouteries Eau de carburant d'hôtel de Taxi de restaurant tout à heure, on va vous proposer, exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi et sorte de grand acte d'enquête quand on demande à quelqu'un, s'il a sa carte de taxi s'il ne l'a pas voir que c'est quelqu'un qui fait qu'il ait pas de taxi, donc oui c'est des délits, monsieur le sénateur, qui sont extrêmement objective able, ils ne demandent pas des recherches d'investigations de police technique et scientifique d'audition et de complexe de complexité qui en en Bolivie, la procédure pénale, quel est le but de notre histoire. Reprenons la belle formule de de Beccaria ce qui compte, c'est pas la sévérité de la peine, c'est sa certitude. Et nous mourrons tous du fait que nous pouvons tant tant qu'on le souhaite, les peines. Si vous n'avez pas la certitude d'avoir cette condamnation et donc la rapidité de ce qu'on a et ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est surtout pour des délits qui nous apparaissent tous mineurs mais qu'il faut quand même pouvoir poursuivre sinon supprimons-les du code pénal, mais le législateur veut qu'on les garde, donc il va falloir qu'on réserve, c'est que cette question : comment on peut avoir des des dit que vous ne voulez pas supprimer dans le code pénal et pour autant qu'ils ne connaissent. Quasiment pas de sanctions, voire pas du tout de sanctions dans la vie réelle, je prenais l'exemple à cette tribune de la consommation de stupéfiants, chacun sait que personne n'était condamné à de la prison ferme pour consommer un joint sur la voie publique et pour autant est-ce que c'est bien de consommer un joint sur la voie publique, nous avons 12 considéré en tout cas, majoritairement qui n'était pas bien, mais il fallait quand même une sanction, avoir des délits sans sanction, c'est comme si, comme disait ma grand-mère, on faisait quelque chose dans un violon et on n'a pas très envie de faire quelque chose dans un violon, on a envie que ce soit on ne peut pas dire, Monsieur le Sénateur, que les délits que nous vous proposons transformée en amende forfaitaire délictuelle soit aujourd'hui particulièrement poursuivi qui donne lieu particulièrement à des sanctions ou à des actes de justice et ils en Bolivie, la vie des commissariats des brigades de gendarmerie et des parquets qui doivent se concentrer sur les délits les plus graves qui en effet mérite des actes d'enquête poussée alors. Là où j'ai du mal à comprendre également le sujet, c'est quand même le le coupé par l'eau du Sénat que accepte de boire le gouvernement, le président de la République a évoqué la généraient sont des AFD pour moins d'un an de prison, c'était un des conclusions du Beauvau, monsieur le sénateur, c'était alors vous dites trois mille deux cents ou quatre cents, nous avons compté avec la DC jusqu'à 3900 délit qui étaient concernés

Les rapporteurs ont évoqué plutôt que des critères une liste, nous sommes passés de 3900 à sept semble-t-il dix bon, vraiment, on peut, on peut discuter mais enfin vraiment, là on est vraiment dans le détail, hein, on en propose quelques autres supplémentaires, le débat va faire naître d'autres propositions, on sera peut-être à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas généraliser que de passer à une vingtaine d'AfD, c'est plutôt une non-généralisation que auquel le procédons aujourd'hui est-ce que ces AFD fonctionne, c'est quand même aussi la grande question qui se pose alors : elle fonctionne. Elle fonctionne en sécurité routière plus personne, pas un gendarme pas un policier ne voudrait revenir à la situation hantée des elles fonctionnent dans la consommation de stupéfiants 260000 AFD mis elle fonctionne différemment selon des types d'infractions, j'ai déjà eu l'occasion de dire au rapport. Avec lui, avait interrogé que l'AFD que vous avez accordée notamment dans la justice de Madame Belloubet l'occupation illicite d'un terrain d'autrui par à certains nombres de moyens motorisés, je n'aurais pas citer ici particulièrement les gens du voyage, mais évidemment c'est de tes l'intention du législateur me semble.-t-il elle fonctionne très moyennement parce que comme il faut reconnaître l'infraction, il est rare que la personne qui s'installe sur un campement illégal le reconnaissent, mais que dit alors le le policier ou le gendarme, si vous ne reconnaissait pas la fraction alors nous allons vous présenter devant le procureur de la République et c'est pas pareil du tout que vous ne reconnaissait pas la fraction, je ne peux rien faire et donc je me retourne dans les élus pour dire bon ben voilà, monsieur, dames, il va falloir prendre votre mal en patience, ou faire une longue procédure, ou peut-être que ces caravanes serait déjà parti. C'est vraiment un outil qui permet le contradictoire et des délits constatés, ainsi qu'une amende qui effectivement est pénal et donc s'inscrit otages et qui permet peut-être aussi de regarder un certain nombre de choses, je prends la consommation de cannabis par exemple ou de cocaïne. à force d'avoir des AFD, on constate que cette personne n'est pas simple consommateur mais et peut être dans un cas d'addictologie particulier qu'il faut évoquer et lorsque le juge a devant lui, quelqu'un qui a eu plusieurs AFD de suite et qui est désormais, il dit ce qu'il vous faut c'est pas simplement une amende c'est vous soignez monsieur, et ça on le sait, pas si auparavant on n'a pas mis les amendes pénales, bien sûr, je terminerai par dire que il y a une petite absence de connaissances totale de l'AFD dans son fonctionnement, comment ça fonctionne, vous allez voter l'AFD, nous allons demander à l'entaille de mettre en place cette AFD, l'AFD va fonctionner le policier va arriver et va constater que vous faites une activité illégale d'exploitant de taxi vous reconnaissez la fraction plutôt que d'aller en garde à vue, vous dites : c'est quand même plutôt sympathique de prendre une amende plutôt que les gardes à vue, c'est ça l'alternative : soit je fais 24 heures ou 48 heures en garde à vue, soit j'ai une amende en général, on choisit d'amende bon. Quand arrive l'amende, je mets l'amende à monsieur X va pouvoir contester la l'amende, évidemment, il ne peut bien évidemment et surtout il y a un 2ème contrôle puisqu'on a fait l'AFD. Selon la circulaire pénale prise par le procureur du territoire qui peut d'ailleurs territorialiser sa réponse pénale par rapport aux dangers que ça représente. Il est certain que l'existence d'exercice illégal de l'activité des taxis sont entrés dans la politique pénale des procureurs, la République et plus grave à Paris qu'elle ne l'est à Tourcoing, j'ai des taxis à Tourcoing, ils font un travail formidable, on peut pas dire que la filouterie à l'exercice illégal de taxi soit le danger 1er de la délinquance tourquennoise, donc on peut dire que là, ce sera plus grave que la si c'est que que que que que dans un autre territoire, donc ça me paraît intelligent commode évidemment de politique. Pénale et puis deuxièmement, il y a un procureur de la République à Rennes, celui qui reçoit tous les AFD mise par les forces de l'ordre qui regardent si c'est AFD, elle est conforme à la circulaire et conforme à la mise en place de ce qu'a voulu le législateur et il y a un certain nombre d'AMD qui saute, arrivée au parquet numérique si j'ose dire, de Rennes, donc vous avez contrairement à d'autres procédures de procureur qui vérifie ce qui se passe le 1er, celui qui fait la circulaire pénale et le deuxième, celui qui regarde. Si les policiers et gendarmes à la fin du CIO ont bien fait cette cette amende ne sont les règles de l'art non vraiment toutes des critiques que vous opposez aux AFD ne me semble-t-il, ne tiennent pas ce qu'il peut tenir, c'est que constater et ce sera l'objet de l'amendement que je vais descendre dans quelques instants, madame la présidente, que telle ou telle délits ne doit pas rentrer dans ce Champ. Soit parce que vous considérez que ce n'est pas un délit facilement objective able donc dans ces cas-là, c'est votre vous soutenez ça monsieur le sénateur, et on peut. Attends, on peut en discussion là-dessus, soit on considère qu'il ne faut pas passer en amende forfaitaire, ce qui est tout ce qui relève de la réponse pénale classique par exemple avec monsieur le rapporteur, nous avons eu un débat pour savoir si nous faisions rentrer les armes comme les armes blanches, le couteau dans une amende pénale ou pas dans une amende pénale, on sait tout ce qu'est aujourd'hui les couteaux pullulent. est très difficile de interdire la vente de couteaux puisque chacun normalement on a chez soi, donc ce serait un peu absurde de rentrer dans un débat comme sur les autres armes : faut-il, pour pouvoir permettre aux policiers, aux gendarmes de réguler le nombre de couteau qui circule dans sur la voie publique le passer en amende forfaitaire délictuelle ou le laisser à la disposition, parce que c'est un acte que l'on peut considérer comme grave devant un d'OPJ et finalement devant un enquêteur, même si on a très peu de réponses pénales, il faut bien l'avouer, sur les porteurs de couteaux qui n'ont commis aucun acte, on peut avoir oublié de ranger son couteau de cuisine, quand on se balade dans la rue, ça peut tout à fait arriver, j'imagine, dans beaucoup de cas, bon, monsieur le rapporteur, ce n'est pas trahir nos secrets que de dire que vous n'étiez pas très favorable à ce que on nous vous proposons une AFD sur ce point, voilà le genre de débat qui est intéressant, c'est pas l'outil AFD qu'il faut combattre, c'est les délits à part, hein, et c'est pour ça, la présidente que je propose qu'on rejette les amendements de à l'article 14 et qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet pour parler délit par délit et notamment ce que j'ai proposé par l'amendement 233. Merci j'monsieur Favreau. ou sur ces délits, vous parlez de délit, celui qui dira j'ai acheté un chien d'attaque et j'avais aucune intention délictuel et moi j'achète un chien il y en a dans toutes les zones d'animalerie, vous allez pas le condamner le tribunal ne le condamnera pas et l'amende forfaitaire sera contestable. Je pense. en vertu de la loi votée par le Parlement aujourd'hui va mettre une amende forfaitaire délictuelle, il me dit : vous n'avez pas le droit d'avoir ce chien d'attaque, je lui dirai : vous avez raison. Et je j'accepte donc puisque je reconnais moi ma réaction : l'amende forfaitaire délictuelle je reconnais donc moins d'infraction.

L'AFD n'est possible que lorsque je reconnais d'infraction et si je dis, moi, je ne connais pas la infraction le policier ne me mets pas d'AfD et donc là, le policier, il a 2 choix : soit. C'est partir avec mon chien d'attaque soit dire bah Monsieur vous aime suivre au commissariat parce que je considère que vous avez fait un délit et je vais vous placé en garde à vue après consulter procure de la République pour appeler votre avocat et contestée devant le tribunal, donc la FED ne pose pas de problème à personne et surtout pas à à au contentieux, que vous évoquez doit tribunaux puisqu'il ne peut pas y en avoir, l'AFD, c'est une forme de peines alternatives, permettez-moi de le dire ainsi, quand je reconnais l'infraction quand je la reconnais pas et que je souhaite rentrer en au contentieux avec l'administration, hé ben dans ces cas-là, je vais présenter mes droits devant le tribunal, donc il me semble que votre argument vient renforcer en fait le mien. Merci, je mets donc aux voix ces quatre amendements avec 2 avis défavorables qui vote pour. Qui vote contre. Qui s'abstient, ils ne sont pas adoptés, Monsieur le Ministre, vous avez largement déjà introduit votre amendement. C'est une l'appel à la concision sinon et neige des présidentielles suivis bien compris, madame la nous proposons la transposition de davantage d'AfD, je rappelle que Monsieur le rapport. A évoqué la filouterie de carburant la filouterie d'hôtel de Taxi de restaurant la violation des règles de Notat pour nos amis routiers les atteintes à la circulation des trains, l'intrusion non autorisée dans une école et les délits en matière de chiens d'attaque, nous venons d'en parler, je propose y rajouter l'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi, je pense que nos amis taxis qui font un travail très important connaissent une concurrence pour le moins malhonnête et donc ainsi nous pourrions répondre à leur demande, l'exploitation de voitures de transport avec chauffeur, son inscription au registre. Chacun ont compris que c'est dans le même, la même circulation routière et de services qui parfois ne sont pas faits sont les règles de l'art, créer une concurrence illégale et ça insécurisait aussi les les personnes qui sont dans ces voitures qui ne. Pas d'information pour la prise en charge un client sur la voie publique pour une prestation de transport sans justification de réservation préalable par une personne ayant pas la qualité de taxi, je pense qu'on a compris que c'était même principe : le refus de se soumettre aux vérifications relatives aux véhicules ou au conducteur la transformation d'un véhicule portant atteinte au dispositif antipollution, le délit d'entrée par force est en état d'ivresse. Dans une enceinte sportive lors d'une manifestation sportive, je suis là, obligé de constater que c'est de plus en plus le cas, notamment dans certains sports et monsieur le rapporteur avait évoqué la dégradation légère dont les tags qui pourrissent la vie de nos concitoyens sont jamais qui devrait sanctions et les dégradations légères avec circonstances aggravantes, voilà madame la présidente, je veux bien avouer devant le Sénat qu'à la lecture de nos débats, le refus de se soumettre aux vérifications relatives aux véhicules et aux conducteurs peut faire l'objet de discussions puisque c'est sans doute celui qui est le moins facile infractions 6 jours aussi, je refuse de donner mes papiers, il faudrait que je reconnaisse aux gendarmes que je refuse de leur donner mes papiers, ça peut arriver, disons que c'est sans doute la FED, la moins efficace par rapport à l'argument qu'a donnée monsieur Favreau mais pour l'instant, je la maintiens, si vous souhaitez un débat dessus aussi, nous en discutons avec l'semaine nationale ou en CMP. Merci monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, votre avis. Un président sans surprise, la, la, l'avis de la commission des des lois et est favorable à cet amendement déposé par le gouvernement, hier, nous avons un débat spécifique à la commission des Lois

amendement du gouvernement, ça permettra d'avoir, sur ces 24 amende forfaitaire délictuelle, une analyse un suivi qui sera concret opérationnel et qui permettra, le cas échéant, d'avoir un avis sur le développement modéré raisonnables de ce type de de sanctions dans les dans les, dans les mois qui viennent, évidemment, la navette, monsieur le Ministre fera son oeuvre, j'imagine que les députés auront peut-être des idées complémentaires ou des, ou des choses à retirer dans cette liste, en tous les cas, je, je trouve que le travail que nous avons pu mener avec le gouvernement sur cette sur cette liste en en resserrant vraiment les AFD aux infractions où elle serait le plus opérationnel et de bon aloi et je j'engage les collègues à adopter cet amendement. Merci, monsieur le rapporteur, je mets donc cet amendement voit avec un avis favorable de la commission qui vote pour. Contre, abstention il était adopté, Monsieur le Ministre, l'amendement 55 Monsieur Bénard Roche. L'amendement 57 qui était destiné en fait à compléter des alinéas de la tienne, l'article 14 par une phrase qui disait l'agent informe systématiquement des droits de recours de l'amende forfaitaire délictuelle

bon, OK, vous savez très bien comment ça peut se passer, y compris, ça m'est arrivé, mais ça peut arriver à beaucoup d'entre nous de se retrouver dans des cas où il peut y avoir une amende, bon, on a tendance naturellement à accepter la mode surtout que dans, dans, dans le cadre, et je parle, c'est tout à fait logique donc, on l'accepte, je comprends très bien qu'il y a des gens qui peuvent avoir des difficultés et qui, même s'il ne devrait pas pour une raison ou pour une autre l'accepter en fait se disent qu'ils ont pas d'autre moyen d'échapper à au passage à la gendarmerie au poste de police à un certain nombre d'heures immobilisé dans leur emploi du temps, y compris s'il travaille et etc, que de l'accepter même si au fait il ne voudrait pas l'accepter, donc moi je dis juste que dans ce cas-là, simplement je pense qu'il faudrait faire en sorte que les forces de l'ordre, enfin les personnes qu'ils qu'qui la mettent cette cette amende forfaitaire préviennent systématiquement en tout cas, que ce soit inscrit qu'il faut qu'ils préviennent systématiquement les intéressés qu'ils peuvent contester ces amendes devant le tribunal de police je ne dis pas qu'il va pas le faire, je dis juste qu'il faut les prévenir, à ce moment-là qu'ils peuvent le faire, c'est tout. Merci, votre avis, monsieur le rapporteur. Alors, puisque madame la présidente, monsieur Ménard Roche nous invite à à être dans le réel, dans la réalité. Sur un avis d'amende, il y a la précision écrites ah vous dites, vous l'avez dit en commission, chers collègues, vous le dites un nouveau qui, ça et ça se passe pas comme ça dans dans la vraie vie, mais dans la vraie vie, sur la vie de l'amende, c'est indiqué. Donc pour moi, cet amendement est est complètement satisfait par la réalité de terrain : avis défavorable. Merci, monsieur le Ministre. Oui, en 20 secondes, comment ça se passe, on vous met n'AUD je ne sais pas si vous avez vu récemment, monsieur le sénateur vous et je ne sais pas de quel type d'ailleurs, je ne veux pas en détail, on met une AFD le policier, gendarme, vous dit vous reconnaissez, vous avez dit oui il vous présente le terminal néo parce que c'est comme ça que ça se passe désormais et vous dit faut signer et il y a un petit. Petit cadran pour dire, en gros, vous avez le droit de, et notamment les mentions qu'on pourrait appeler les mentions du contrat émotion qui expliquent que, effectivement, vous avez tout à fait le droit de contester, bien sûr, donc c'est déjà le cas, je vous invite à vous rapprocher de forces de police et de gendarmerie vous, il peut vous montrer comment ils mettent les les AFD vous devez signer, hein, c'est quelque chose de positif, vous devez faire un acte et vous avez tout à fait le droit de constater les choses avant, donc il me semble très satisfait. Monsieur Bernard Roche pour expliquer, explications de vote, sans rentrer dans le détail de votre vie privée. Non, je veux pas rentrer dans le détail des bancs, juste une chose : oui, bien sûr, c'est écrit dans un petit carré sur un écran, OK, on est, on je lui dis ça, excusez-moi, il vous échappera pas : qu'y a un certain nombre de personnes l'oralité n'est pas l'écriture, on sait pas forcément lire ou écouter une parole de la même façon, il y a des gens qui comprennent pas forcément ce qui est écrit en français, quelque part, il y a des gens qui ne savent pas forcément lire il y a, il y a des tas de raisons qu'il faut que, simplement, je ne comprends pas pourquoi le fait de le dire, en plus de fait qu'il soit écrit sur un petit bout de pages ou de feuilles ou d'écran poserait un problème. Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui votent pour, contre, abstention, il n'est pas, z'monsieur le rapporteur pour la commission des lois, l'amendement oui parfait je mets donc aux voix cet amendement avec l'avis favorable du gouvernement qui votent pour, contre, abstention il était adopté, monsieur Richard, l'amendement 209. Ils ont autant pour moi je j'ai pleinement approuvé la démarche de la commission, et ensuite celle du gouvernement par son nouvel amendement de recadrer

en mentionnant parmi les les fêtes justiciable de d'une amende forfaitaire, le port d'arme, c'est d'une arme blanche, il peut s'agir de la la catégorie D c'est-à-dire poignard matraque point électrique ou carabine à air comprimé, comme le ministre l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'un phénomène qui est en propagation qui en n'extension qui porte par lui-même dit danger et qui est assez souvent le vecteur d'attitude, de menaces ou de pression dans la vie interpersonnelle, il me semble donc que je reste enfin cette propositions reste dans la cohérence de la démarche qui a été celle de la commission du Sénat dans ses votes antérieurs en limitant l'usage de cette procédure particulière à aisément objective able et présentant une atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, j'insiste donc pour que nous inclusion le port de ces armes dans les actes justiciables de l'amende forfaitaire. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît.

à la fin de l'année, au profit d'un nouveau dispositif, et au regard de la recrudescence des attaques à l'arme blanche, il convient de de s'interroger sur le caractère adéquat de la réponse pénale pour nous, c'est plutôt un avis défavorable à l'extension aux armes de de au port des armes de catégorie D. Monsieur le Ministre, en garde à vue, tout le monde en procédure pénale parce qu'on porte un couteau ou une matraque sur soi alors que les choses pullulent, je rappelle d'ailleurs que les dernières attentats terroristes ont tous été commis avec ce genre d'armes et non pas avec des armes plus complexes, donc je suis favorable à un moment sur Richard. Je mets donc aux voix cet amendement avec un avis défavorable de la commission favorable du gouvernement qui vote pour. Qui s'abstient, il n'est pas adopté. Monsieur Richard, l'amendement 210.

de l'amende forfaitaire éteint la procédure pénale, or il peut y avoir un dommage qui a été créé à une tierce personne, une victime par le l'auteur défaite et donc ce que ce que ce que souhaite cet amendement c'est de compléter : j'ai un point le code de procédure pénale, en précisant que lorsque le délit a donné lieu une amende forfaitaire ça ne ça ne prive pas la victime, les victimes de demander au procureur de la République de citer l'auteur devant le tribunal pour que soit statué sur les intérêts civils, c'est-à-dire sur le préjudice de la victime. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Cette mesure préserve les droits des parties civiles et nous est apparu totalement opportune l'avis de la commission des lois favorable. Monsieur Miss favorable je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis favorable qui vote pour. pour. Abstention il être adopté l'amendement 213 Madame Darcos. Merci madame la présidente, cette cet amendement de de ma collègue elle Joseph et et signée par beaucoup d'entre nous, il a pour objet de reprend le dispositif proposé par la proposition de loi qu'elle avait déposé le 30 mars 2022 afin de mieux lutter contre les infractions en matière d'urbanisme, par le biais d'une amende forfaitaire, en effet, pour améliorer l'efficacité des procès-verbaux dressés par les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, la proposition de loi suggère d'instituer la possibilité de prononcer une amende forfaitaire délictuelle pour tout procès-verbal qui infligerait une amende dont le montant pourrait aller jusqu'à 3000 euros dans les infractions mentionnées au 3ème alinéa de l'Arctique L 481 tirer 1 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire celles prévues par les articles L. 480 tiré quatre il s'agit des travaux effectués en méconnaissance des articles L. 421 tirer hein, ah elle 421 tiré 5 du code de l'urbanisme, cela vise des constructions sans permis de construire les travaux installation aménagement sans permis d'aménager ainsi que les démolitions de constructions existantes sont permis de démolir en effet infractions au code de l'urbanisme constitue surtout un certain nombre de CD dix pourrait donc être puni d'une amende allant jusqu'à 3000 euros est ainsi proposé de prévoir l'application de ces dispositions du code de procédure pénale qui rendent possible le recours de l'amende forfaitaire, conformément à ses dispositions qui renvoie à l'article 131 tiré 13 du code pénal : l'amende forfaitaire délictuelle ne peut excéder un montant de 3000 euros, il sera donc possible d'infliger une amende forfaitaire pour tout délit pouvant donner lieu à une amende de 3000 euros

en indiquant que l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire le paiement de l'amende forfaitaire mettrait fin à l'action publique, donc la procédure pénale par un procédé qui serait non seulement répressif mais dissuasif. Mes chers collègues, monsieur le rapporteur, votre avis. Alors vous êtes ici au Sénat dans la chambre, qui représente les collectivités locales n'emmène notamment les maires sur le fond, cet amendement pose une vraie difficulté législative logistique c'est que elle, elle ne fixe pas un montant forfaitaire mais elle dit jusqu'à et donc ça n'est pas ce que nous avons dans les 24 désormais 24 autres AFD voter les dix existantes et les 14 que le Sénat a adopté, donc ça ça pose une vraie difficulté et j'attire votre attention, mes chers collègues, sur une autre dimension, c'est que le maire est OPJ que le maire délivre audits de son pouvoir de police administrative des autorisations d'urbanisme que c'est en contradiction à ces autorisations d'urbanisme, ce que un certain nombre de contrats de de construction pourrait être considéré comme illégal et si on donne à la même autorité de, de, de délivrer des autorisations d'urbanisme, si cette même autorité et exerce vous dites d'un autre pouvoir de police des pouvoirs de police judiciaire, il y a une espèce de conflit. D'intérêt au de, de, de mission entre entre les deux et et honnêtement, autant on est tous pour le renforcement des pouvoirs des maires, tous pour le fait de de conso de considérer que beaucoup de de ces problèmes sont des problèmes lourds. J'ai été maire pendant 10 ans, je sais de quoi je parle, j'ai, j'ai vu des choses très concrètes et on est très nombreux ici à avoir exercé ces fonctions-là, mais de là à donner au maire. Un carnet à souches ou un terminal mobile pour délivrer des AFD sur des constructions illicites en qui vont à l'encontre d'autorisations qui ont été données, ou qui n'ont pas été donné par la même autorité, je pense que on s'aventure sur un un terrain extrêmement glissant, ne donnons pas des pouvoirs à nos mères qui sont des pouvoir de shérifs, sauf à les engager à avoir de vraies difficultés sur un plan juridictionnel, par la suite, donc c'est un une demande madame la sénatrice, chers collègues de retrait pour être retravaillé, peut-être dans un autre cadre. Monsieur le Ministre. Même avis. Monsieur le le président. La collègue qui a défendu cet amendement et celle qu'il a élaboré qu'il aurait fallu aller un tout petit peu plus loin dans le code, parce que nous avons adopté il y a plusieurs années, un article L 481 tirer, hein, qui prévoit des moyens de pression administrative à la à la possibilité du maire dans la continuité de son pouvoir, délivrance du permis, c'est-à-dire qu'il peut imposer une consignation à la personne qui est en infraction permis pour qu'elle fasse les travaux de remise en état et il peut lui imposer une astreinte simplement au moment de la liquidation de l'astreinte, ce sera sous contrôle du tribunal.

en fait, c'est sur les AMD et le Conseil d'État, on en a parlé tout à l'heure, il soulignait, en fait, l'absence d'évaluation préalable bon s'agissant des contentieux relatif à l'usage des stupéfiants, je l'ai dit tout à l'heure, on peut considérer effectivement que c'eût été utile de faire maintenant une évaluation a posteriori par exemple, c'est, c'est la raison pour laquelle des syndicats et des associations de professionnels de la justice ont demandé s'il n'était pas possible, en fait, et nous ne

et fiction dans la loi, la date limite à laquelle nous devra l'évaluer voilà. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Madame la présidente, en réponse à notre collègue Guy Bénard Roche et à cet amendement, d'abord on a refusé la généralisation. Donc ça veut dire que l'évaluation que vous proposez, elle porte sur 20 24 infraction pénale. J'ai la certitude et je me permet de penser que j'ai quasiment la garantie de la part du ministre que à chaque fois qu'un parlementaire demandera la communication des chiffres José 24 infraction le gouvernement quel qu'il soit répondra à cette question là et on n'est pas du tout sur une une réforme de l'ampleur que c'est celle qui était envisagée au départ et que, en fait, en plus de ça, c'est même pas sur les 24 infraction qui avait que qu'il y aura des questions mais sur l'une ou l'autre, et à ce moment-là,

Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour. Contre, abstention, il n'est pas adopté, j'ai mis aux voix, l'article 14 modifiée qui votent pour, contre, abstention il être adopté, nous avons des articles additionnels après l'article 14.

le maire et les adjoints ont le pouvoir de constater et de verbaliser eux-mêmes les contraventions susceptibles d'être sanctionné par le système de l'amende forfaitaire, le recours à ce dispositif est toutefois rare car les maires n'ont bien souvent pas connaissance de cette possibilité des différentes infractions qui peuvent être sanctionnés de la procédure à suivre, par ailleurs, cette procédure se heurte à un obstacle pratique l'approvisionnement en carnet à souches n'étant, semble-t-il, pas sans difficulté nombre d'imprimerie, nous n'en produisons plus les communes ne dispose malheureusement pas pas non plus des outils permettant le relevé de l'amende forfaitaire par procès-verbal électronique qui représentent un coût non négligeable pour les plus petites d'entre elles, alors que ce dispositif se généralise en l'absence de police municipale et avec la disparition des garde-champêtre, certains maires souhaiterait pouvoir recourir à ce dispositif, il conviendrait d'améliorer l'information des mères et de leurs adjoints sur leurs pouvoirs en matière de verbalisation les infractions concernées et les modalités à respecter le présent amendement prévoit également d'expliciter dans la loi ce pouvoir de verbalisation des mers. Si monsieur le président, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Oui, l'amendement, madame la présidente du du du de notre collègue Hervé Maurey, présenté par Laurent Lafon, permet d'avoir un débat très intéressant. Sur la question des pouvoirs de police du maire, le fait que nos, nos collègues maires sur le terrain, dans les 35000 communes de France, hé bien conscience de l'étendue de leurs pouvoirs de police administrative d'une part de l'étendue de leur de, de, de leur pouvoir en matière de police judiciaire, d'autre part, étant précisé qu'ne pourra pas faire un colloque juridique sur la le fait de savoir si les prérogatives

à la police municipale qui doivent devrait l'exercer en propre et que s'il l'exerçait en propre, ils encouraient évidemment toute la responsabilité que cela recouvre et on a parlé longuement de la formation des OPJ en début d'après-midi. Cité l'été le cas, il faudrait que les maires se soumettent à la même formation que les OPJ policiers nationaux ou gendarmes pour être en capacité sur le terrain de délivré effectivement ces ces amendes forfaitaires délictuelles l'amendement de d'Hervé Maurey, à mon avis, permet de Lens d'enclencher un débat, je ne suis pas sûr qu'il apporte la réponse tout à fait idoine qu'il qu'il enclenche et c'est la raison pour laquelle la commission des lois a souhaité connaître l'avis du gouvernement, sur une question aussi sensible que l'étendue des pouvoirs de police judiciaire du maire dans la réalité du terrain actuellement en France. Monsieur le Ministre votre avis donc. je suis défavorable à cet amendement, mais pas pour les mêmes raisons, c'est qu'il me semble que le maire étant un officier de paix judiciaire certes originale, mais officier policière, judiciaire quand même peut émettre des contraventions et même des amendes forfaitaires délictuelles, à partir du moment où un certain nombre de règles de droit qui sont. Propres aux élus soir sont respectées, ils ne font bien souvent à travers leurs services municipaux et notamment leur police municipale mais il peut le faire directement, ça m'est arrivé, lorsque j'étais moi-même maire mais il est évident que il faut davantage encadrer ce droit d'abord pour le rendre plus lisible de la part des élus locaux et je veux bien avouer que notamment les maires des communes les plus petites de France sont souvent un peu ignorant de la façon dont ils peuvent adresser ses contraventions, ce qui, nous, on a par exemple pas de garde-champêtre, pas de policiers municipaux qui, d'habitude, on la délégation de ce pouvoir du maire, et par ailleurs, je veux bien aussi remarquer que les procureurs ne suivent pas toujours les contraventions ou les demandes des maires encadré dans un OPJ 10 particulier. Il me semble, en tout cas que c'était pas la place dans ce texte de revoir le pouvoir de PJ du maire qui pose bien d'autres questions et notamment celle de la chaîne pénale ou de ses pouvoirs propres au code général des collectivités territoriales, ce que je proposerai à monsieur le président de la commission des lois, puisque beaucoup d'entre vous m'envoie sont souvent leurs documents de sénateurs et j'ai notamment vu que ah, sénateur de ma propre région, je pense au sénateur Demilly, il a fait passer d'envoyer ça il y a quelques jours un petit document avec notamment trois quatre pages sur les pouvoirs d'OPJ du maire et les contraventions, comment on fait une contravention sa de son département, je, je dis ça pour les uns et les autres et et aura ainsi dire la la version simplifiée du bon sens que de Stéphane Dominique je connais depuis très longtemps, j'avoue moi-même que si j'avais été maire, je me serais posé des questions sur plus à la fin qu'au début de sa propre présentation alors des gendarmes essayent souvent dans les communes rurales de faire des formations spécifiques, j'espère qu'ils le font, je sais que prison la fronde relève pas toujours d'un département qui est propre à la gendarmerie nationale, mais je croyais qu'ils le font, là où ils peuvent le faire, c'est vrai que les policiers ne le font pas, et ça je pense que c'est un un problème parce qu'en zone urbaine, on peut être confronté évidemment même problème en tout cas moi je suis prêt Monsieur Président maintenant qu'une partie des collectivités locales et et notamment sur la compétence, c'est que la DGCL très rapidement, pourquoi pas, dans un texte qui pourrait relever soit de du garde des Sceaux, soit un texte propre à la sécurité, vous savez qu'on en aura d'autres très bientôt, soit une promotion. On doit évidemment sénatoriale a travaillé en parfaite Intelligence pour clarifier l'OPJ mère qui n'est pas tout à fait bien compris par chacune et par chacun et parfois par les propres services de l'État, donc un avis plutôt de retrait. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis donc. Oui, à la lumière de des des informations et et des et des éléments de réflexion, porté par le ministre, nous nous rangeons l'avis du Gouvernement demandant le retrait de cet amendement. Monsieur le président vous retirer. Tenu des des arguments avancés par le ministre et surtout de cette ouverture au dialogue sur ce thème important pour le maire, je je vais retirer l'amendement. Merci monsieur le président, nous passons à l'article 14 bis, avec une demande de prise de parole de monsieur Bena Roche. Merci madame la présidente, en fait, cette prise de parole à à pour but essentiellement de rappelés 3 choses : la première c'est que nous avons un certain nombre d'amendements qui ont été déclarés recevables comme certaines de nos confrères d'ailleurs une dizaine dans dans cinq, qui porte sur les articles 14 bis et quinze sans que nous ayons vraiment compris totalement mais je suis sûr qu'il aurait été à juste titre, mais en tout cas on n'a pas compris forcément totalement la cohérence des amendements qui étaient recevables par rapport à d'autres en fonction des des différents débats et textes de loi qui a eu et et propositions de loi, enfin, amendement qui a été fait ici, bon, je regrette, entre autres, par exemple du de ce fait que nous ayons pas pu débat du port d'arme des policiers hors service dans les ERP qui était quelque chose dont nous avons discuté, oui d'accord mais on pourra discuter dans ce cas de là aussi parce que, alors j'en arrive à la 2ème remarque parce que je vois, Loïc Hervé qui me presse il a raison d'ailleurs parce que leur tourne sur ce. Sujet : que nous dit le ministre, en fait, le ministre nous dit et il a raison, je suis d'accord le ministère doit nouer des Liens avec la recherche et les études semblent nous montrer Monsieur le Ministre, peut-être en avez-vous d'autres je ne sais pas qu'avec l'augmentation du port d'armes, y compris dans l'ostensible les violences augmentent de près de 15 ou bien encore que plus d'attaques armées aurait été déjoué, sans l'aide de riposte armée qu'avec alors il y a sûrement d'un chiffre qui disent des choses, pas tout à fait les mêmes parce que je veux dire c'est que le débat est ouvert et il nécessite au moins de pouvoir avoir des des études et et de pouvoir en rediscuter et remettre le métier sur l'ouvrage, une nouvelle fois, nous aurions aimé pouvoir discuter de mesures dont nous pensons qu'elles n'ont pas été prises dans une réflexion apaisée, nous faisons également part de quelque chose qui nous a semblé peu cohérent des fois d'ailleurs pas de la part du ministère mais de la part de, de, de, des rapporteurs ou ou de l'hémicycle en est du souvent on en a discuté, on en a décidé, alors peut-être que la nouvelle règle maintenant, c'est de dire : on ne peut pas discuter de foi des mêmes sujets, on en a discuté, on en a décidé, on ne peut pas rediscuté je m'adresse pas à vous, Monsieur le Ministre, là je m'adresse à avec Oleg, bon c'est pas ce que c'est pas ce qu'on pense, mais dans ce cas-là, pourquoi, pourquoi traiter de la réforme de la des PPM avant l'arrivée du rapport d'ailleurs, on nous l'a souvent dit, on va pas traiter de l'information, on va pas traiter, il y a plusieurs sujets dans le rapporteur de Brest nous a dit : ben, on va pas les traiter matelas puisqu'il y a un rapport qui arrive, OK, mais donc dans ce cas-là on il y a, il y a quand même une une incohérence deux où on les traite de fois où on fait le rapport avant et on les traite quand même voilà donc tout ça nous a un peu perturbé dans cette façon d'étudier la loi et comme mon temps de parole partie je m'arrêterai là. cher collègue, nous passons l'amendement quarante. Du hein monsieur le Président, sueur parfait. Nous allons voter sur l'article 14 bis qui vote pour, contre, abstention bah, écoutez, dans l'indifférence générale, l'article 14 s'est quand même passé nous allons étudier maintenant les articles additionnels après la a-t-il 14 bis Madame Noël. Oui, c'est ça Madame Noël pardon votre amendement numéro 127. Merci madame la présidente, monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes nombreux dans cet hémicycle à subir les occupations illicites de gens du voyage et mon département, de la Haute-Savoie est particulièrement concerné par cette question, mais je vais aujourd'hui vous parlez d'un tout autre phénomène à travers cet amendement, je souhaite mes chers collègues vous sensibiliser sur les agissements répétés de groupes qu'on a encore du mal à qualifier de gens du voyage tentent ne voyagent plus ou très peu et s'apparente davantage à des voyous sans foi ni loi qui ne respectent rien, se moque de tous les sans-à chacun de leur passage une désolation une colère immense aire saccagée détérioré activité entravée délits en tout genre, chaque année, les situations se répètent et ne manque pas de susciter l'exaspération des élus et de nos concitoyens et pourtant malgré ses méfaits ces communautés peuvent continuer à se prévaloir des dispositions de la loi Besson qui prive la collectivité de pouvoir bénéficier de l'expulsion par la voie administrative, c'est-à-dire la plus rapide, la moins coûteuse et la plus efficace dans l'hypothèse où cette même collectivité n'aurait pas complètement rempli ses obligations au regard du schéma départemental d'accueil des gens du voyage schémas toujours plus exigeants, coûteux et dont les dispositions ne sont plus tenables pour les élus cela n'est plus l'admissible, la loi Besson entre chaque jour ses limites et ses failles qui conduisent à de telles dérives instaurant beaucoup de droit pour chaque pour certains et beaucoup d'obligations pour d'autres, lorsqu'une commune ne remplit pas totalement ses obligations, elle ne peut que recourir à une procédure judiciaire fastidieuse, longue coûteuse et attendre parfois plusieurs semaines pour voir la force publique, faire exécuter cette décision, laissant ainsi tout le loisir à ces groupes de prolonger leur séjour irrégulier, parfois pendant plusieurs mois sans être inquiété le déséquilibre des droits et des devoirs de chacun épatant et je vous propose, à travers cet amendement de corriger cette cette injustice au bénéfice de nos collectivités locales et de nos concitoyens qui ne peuvent plus tolérer ces amendements mon amendement propose donc que les communautés qui se sont rendus coupables d'agissements direct UE ne puisse plus se prévaloir des dispositions de la loi Besson et que l'on puisse, dans tous les cas, mettre en oeuvre la procédure administrative pour les expulser, je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, votre avis s'il vous plaît. Oui, madame la présidente, bon Madame Noël et les nombreux collègues qui ont signé cet amendement savent combien je partage la préoccupation de faire progresser la question des installations illicite des, des, des gens, des gens du voyage, alors cet amendement, il pose de difficulté : la première c'est qu'ils suppriment une amende forfaitaire délictuelle, qui n'est rentré en vigueur qu'au mois de janvier 2022, bien que le Sénat les voter la fin de l'année 2018 on nous avons bataillé de haute lutte pour que cette AFD soit mises en place cette AFDL pose des très très grandes difficultés sur le terrain puisqu'elle suppose la reconnaissance de l'infraction par la personne qui est mise en cause et en elle est en réalité cette reconnaissance de la, de l'infraction n'a n'intervient quasiment jamais et il faudrait que des consignes très claires soit données aux forces de police et de gendarmerie pour que, dans la mesure où cette AFD ne peut pas être mise en oeuvre du fait de la non-reconnaissance de l'infraction que il y a une prise en charge au titre de la flagrance otite de la gravité du délit qui commis quand même pour qu'une réponse pénale soit à apporter rapidement sur le terrain et d'ailleurs, indépendamment des questions de conformité ou pas au schéma départemental tant le schéma départemental et difficile à obtenir dans un territoire frontalier comme le nôtre et et malgré la bonne volonté des élus d'y parvenir donc une vraiment une monsieur le ministre, une question sur cette AFD pour qu'elle qu'elle puisse être, elle est en plus une mise en mise en oeuvre de manière différenciée suivant les les parquets, donc on est vraiment une espèce de doctrine qui soit mis en en hausse sur cette sur ma chère collègue c'est un c'est un un sujet qui touche à la loi Besson, son application, alors là, ça dépasse complètement, on le, je l'ai dit à plusieurs reprises dans le texte, ça dépasse complètement le le le périmètre du texte, nous n'avons mené aucune audition avec ma fille, Daubresse sur la question, profs, des gens du voyage je botte pas en touche, mais je pense quand même que sur sur ces questions-là, il faut vraiment que nous avancions mais je suis pas sûr que cet après-midi, ce soit exactement le le bon endroit l'avis est défavorable plus plutôt une demande de retrait. Monsieur le Ministre votre avis. Oui merci me monsieur le rapporteur, mais moi j'ai compris de votre amendement madame la sénatrice que vous ne remettait pas en cause en soit la la maison même si j'ai bien compris que vous aviez des questions autour de sa légitimité et, en tout cas de son application mais vous dites un groupe qui, même sur un terrain public dont ils ont le droit d'occuper parce qu'il y a la commune n'a pas à accepter le schéma voulue par le président du département, en tout cas par l'organe délibérative du département ne puisse pas s'installer, s'ils ont commis des infractions, c'est ce que j'ai compris de votre amendement, ça me paraît intéressant puisque la loi Besson dans sa philosophie, c'est l'accueil des gens du voyage, ce n'est pas à l'accueil absolue de toute personne qui commet des actes délictuels qui viennent aggraver le bien public qui transforme leurs droits, pour lequel on accueille des gens dans dans des conditions évidemment de violences et de dégradations sans jamais payer des de ces réparations ayant été maire je vois parfaitement ce que vous souhaitez dire la petite difficulté de votre un moment que je peux accepter sur le principe, c'est que vous évoquez le groupe. Et que je ne vois pas comment, sauf à faire de la du plaisir démagogique je puisse, en tant que ministre de l'Intérieur évoquait que dans le code pénal, on puisse évoquer un groupe sans définir lequel et ce groupe pourrait peut-être même changer parce qu'on pourrait imaginer que sur les 15 ou 20 personnes qui sont là et qui reviendrait cinq six ont même changé et à coup sûr. D'abord le conseil chez à mon avis il va censurer parce qu'on ne peut pas faire en en pénale selon la faute d'autrui, mais par ailleurs, pour le coup, la procédure serait très largement remise en cause, sans doute par la partie des fondante en expliquant que sur les 20 qui sont revenus, certes quinze ont peut-être été confondu de ces dégradations mais qui était nouveau et on ne pourrait pas priver leur droit à eux si vous voulez, ce que je veux dire, donc si je comprends un dispositif que. C'était mettre en place, je pense, mais c'est normal parce que le droit est complexe et surtout s'il est pas passé en commission, que ça ne vole pas, comme disent les techniciens en général pour dire que l'amendement ne peut pas être considéré comme acceptable et et comme produisant des effets qui correspondent à votre demande, ce qui est certain, peut être, monsieur le rapporteur, et monsieur le président de la commission des des lois, c'est que, avec les occupations de caravanes sur les terrains, nous avons un sujet, alors nous on a un triple sujet je voudrais rappeler ici et je crois que je parle à 2, sénateur de Haute-Savoie, si j'ai bien compris vos Terres d'élection, d'abord je voudrais rappeler ici que il appartient au conseil départemental d'élaborer un schéma et que, ayant été conseil départemental moi aussi il faut parfois prendre ses responsabilités et que ces schémas peuvent comprendre qu'il y a ici trop d'urbanisation là une frontière là fleuve là des difficultés que la loi SRU, par exemple, et que on, on doit pouvoir lorsque des communes ne peuvent pas recourir à la force publique parce que elles ne sont pas conformes au schéma départemental avant de demander le changement de la loi, où l'intervention du préfet, peut être que les élus départementaux pourrait dessiner un autre schéma c'est ce que j'ai fait dans mon département, mais chacun peut constater, je ne dis pas que tout est absolument parfait dans le département du Nord, qui voit aussi passer beaucoup de, de, de, de gens du voyage dans des conditions qui ne peuvent pas être difficile pour eux comme pour la puissance publique, les choses se sont beaucoup calmé pour les communes en acceptant par exemple que plusieurs communes puissent mutualiser ensemble une aire d'accueil des gens du voyage, c'est pas seulement ce que j'ai fait dans ma propre. Commune avec d'autres communes qui étaient dans la même situation, mais pour cela, j'ai obtenu avec la majorité départementale, un changement du schéma, donc je crois qu'on savoir puisque je comprends bien, et je lis la presse et je suis au département, il n'y a pas extrêmement longtemps la première des choses serait sans doute que le conseil départemental et je salue par avance le président ça puisse refaire le schéma d'accueil, les services de la préfecture de Haute-Savoie sont à votre disposition pour vous accompagner dans leurs ce schéma. Deuxièmement, la question se pose de l'applicabilité désormais de la loi Besson, et notamment de la loi Besson de avec les autres contraintes qu'on ne fait imposer aux élus locaux, je pense notamment à la loi SRU. Personnellement, je sors de mes capacités, le ministre de l'Intérieur, mais je veux le dire à l'ensemble des collectivités, puisqu'à la fin c'est intérieurs qu'on vient chercher pour expulser les personnes par au cours de la force publique, il apparaît un peu. Inopérant que de dire à une commune qui peut être à peu de foncier qu'elle doit à la fois atteindre la loi SRU et atteindre une aire d'accueil des gens du voyage et il peut y avoir un conflit d'usage, moi je suis pour, je sais que le gouvernement lui-même n'a pas été très positif dans cette question, mais je pense que la Haute Assemblée. Pour le pousser, ça me paraît le bon sens, que ceux qui font une aire d'accueil des gens du voyage puissent se voir diminuer l'obligation de la loi SRU, parce que c'est une forme aussi de l'argent. Social, pas toujours, mais enfin quand même, on voit bien de quoi on parle, parce qu'il faut scolariser des enfants parce qu'il faut ramasser des ordures parce qu'il faut faire les équipes, les équipements électroniques ou électricité si vous ne on a accepté que la loi SRU serait diminuée d'autant, parce qu'on a fait des places d'accueil des gens du voyage, les schémas départementaux serait plus facile à faire, vous les respecterions d'avant. Et donc vous seriez mieux plus fondés à demander l'expulsion des des du terrain et donc le préfet pourrait vous les accorder, troisièmement, je veux aussi souligner la grande difficulté qu'il a à voir plusieurs propriétaires publics ou privés, alors quand ces propriétaires privés et que par ailleurs ils ne portent pas plainte parce qu'on ne retrouve pas, par exemple, le proprio. C'est-à-dire de ce terrain dans ma propre commune, il y avait des Terres industriels, on sait même plus à qu'ils appartenaient parce qu'ils ont été abandonnés pendant 30 ou 40 ans, c'est les mêmes désagréments pour tout le monde sauf que c'est sur un terrain privé et tant que l'auteur du terrain privé ne porte pas plainte, on ne peut pas porter plainte à sa place, et donc nous subissons ces désagréments, on confond souvent au terrain privé et désagréments publics, il faut sans doute que le législateur, monsieur le rapporteur. Se penche sur cette question et peut-être permettre à la puissance publique de se substituer au bout d'un certain temps à la non, plainte déposée par le propriétaire du terrain et il m'est aussi arrivé de constater qu'il y a plusieurs terrains publics sur la parcelle où les gens se sont constatés et si le département n'est pas d'accord avec l'intercommunalité qui est pas d'accord avec le syndicat qui est pas d'accord avec la commune, on ne peut pas expulser des personnes, ce que je veux vous dire madame la sénatrice, c'est que derrière le fait que vous, vous l'avez dit, et je l'entends souvent le préfet refuse de recours à la force publique, parfois, il le fait passer. Qu'il oublie de regarder sa boîte Mail vous répond pas toujours à son téléphone dans ces cas-là, n'hésitez pas appeler, ministre de l'Intérieur, comme le fait Monsieur Hervé, je crois que tous les, tous les, tous les parlementaires, mon portable et sinon prenez-le bien volontiers, il arrive que parfois les préfets ne fassent pas tout à fait, ce qui devrait faire, mais dans l'immense majorité quand je vérifie les cas qu'on me donne, c'est que le terrain est privé ou que l'un des que l'un des propriétaires du terrain public ne s'est pas mis d'accord avec son voisin ou que le maire n'est pas conforme au schéma départemental parce que le schéma départemental n'a pas été revu depuis très longtemps, c'est très compliqué de faire un schéma départemental de gens du voyage surtout la veille des sénatoriales, je veux bien l'admettre ou la veille des municipales mais personnellement, je l'ai fait, finalement, on s'en sort plutôt bien, et surtout, c'est toujours mieux pour l'ensemble des habitants de voir qu'on peut être conforme à la loi, je veux aussi dire qu'il y a aussi plein de gens du voyage qui s'installe, qui vivent du fruit de leur travail, qu'ils avaient worked leurs enfants, la République a reconnu qu'ils avaient le droit de vivre ainsi, il faut désormais qu'on adapte la loi aux difficultés que nous on connaît essayer, c'est parce que vous avez fait madame un peu ce que je vous ai dit que j'étais d'accord ce principe essayer d'encadrer plutôt nos pratiques plutôt que de crier. Donc

un débat qui est un pas important qui n'est pas d'ailleurs un débat qui ne qui concerne que la Haute-Savoie mais il concerne bien des territoires sur sur le territoire national et qui préoccupe beaucoup les élus sur le terrain, monsieur le Ministre, vous avez raison, que le président du conseil départemental, a un rôle à jouer, mais c'est une double signature. Celui qui cosigne c'est le préfet, donc dans des départements, peut être qu'il faut imaginer qu'à à à mi-vie d'un schéma départemental, il peut être intéressant d'en prescrire la révision pour que les objectifs soient soutenables, je ne parle pas du tout de de réduire l'ambition des schémas départementaux mais qu'il soit simplement soutenable quand vous avez des des territoires, je pense à une agglomération aux frontières de Genève, où vous demandez 45 logements de sédentarisation, vous imaginez ce que ça représente, Annemasse, de faire ce type de projet, monsieur le ministre, on a rencontré le président de la République qui est venu régulièrement récemment dans notre département y vient parfois il a pris devant les parlementaires du département, l'engagement qu'un nouveau texte puisse être étudiée au Parlement, il il y a, il y est favorable, vous avez confirmé cette intention, j'ai presque envie avec Sylvia de Noël c'est le permet de saisir la balle au bond et de vous dire que, alors que nous avons déjà dans les travaux du Sénat, un certain nombre de propositions à faire, nous pourrions les les compléter et assez vite proposer un nouveau texte de loi dans le cadre de de des niches, des groupes de la majorité sénatoriale pour qu'on puisse aller vite et de l'avant, corriger cette amende forfaitaire délictuelle, s'il y a du lieu d'être, en tout cas permettent d'apporter des réponses très concrètes aux élus qui n'en peuvent plus de cette situation, merci Monsieur le Ministre, pour votre écoute et je maintiens, évidemment, la demande de retrait auprès de Madame Dole. Madame Darcos attendez-vous retirer. D'accord madame Darcos, mais merci en fait j'ai cosigné, en effet, l'amendement de de de ma collègue je je verrai ce qu'elle veut faire, mais je voulais également vous dire Monsieur le Ministre, que au-delà des expulsions, moi je je stigmatise pas, en effet, il y a des gens du voyage qui sont bien établies et et qui, et qui respecte les lieux et dans lequel ils sont accueillis, moi je voudrais dire que au-delà des expulsions, après il y a tout ce qui reste sur le terrain, moi j'ai des communes dans dans mon département de l'Essonne, on est aussi très très visitée avec des immondices et des détritus épouvantable, j'ai une ville j'plomb qui va, jusqu', qui a été jusqu'à 22 camp illicite sur sa petite commune et avec vraiment enfin des immondices épouvantable, ils ne savent pas quoi en faire et l'État également et totalement démunis de devant ça, on se retrouve avec des tas, c'est pas simplement des ordures, hein, il y a des choses sûrement très dangereuse et donc on parle beaucoup développement durable actuellement mais il y a également cet aspect-là qui n'est, à mon avis pas assez traité dans les textes et je prends la balle au vont de mon collègue Loïc Hervé je pense que même sur ces sujets-là, au-delà même de l'occupation des terrains, il y a également tout l'après, qui est épouvantable, qui est à la charge des communes et les et les habitants n'en peuvent plus. Merci madame Noël. Oui merci madame la présidente, monsieur le Ministre, j'ai bien compris que mon amendement était un parfait d'un point de vue juridique et et je vais donc le retirer mais mais je suis heureuse qu'on est, on est quand même ce débat puisque, comme l'a rappelé mon mon collègue c'est un c'est une problématique qui est majeur, les élus sont extrêmement dépourvu, il manque aussi de crédibilité aux yeux de leurs populations qui ne comprennent pas pourquoi des groupements qui commettent de tels actes puissent rester des semaines de façon impunie sur des terrains parce que ils doivent recourir à des procédures trop longues, donc je pense que ça, il faut vraiment arriver à à ajuster notre réglementation et évidemment, je saisis le le la l'invitation de mon collègue Loïc Hervé pour vous inviter à venir rencontrer les élus de Haute-Savoie, qu'on puisse exactement vous exposer les difficultés qu'on rencontre au quotidien et qu'on puisse envisager une évolution de la loi Besson et puis sur les aires d'accueil pour pouvoir les décompter des obligations de la loi SRU, hé bien sachez que ça a été une de nos demandes à plusieurs reprises et demande qui a toujours été rejeté par votre gouvernement, qu'on trouvera un jour un compromis sur cette question qui, sur laquelle on est également très attendu, je vous remercie. Merci monsieur Roche pour une demande de rapport votre amendement 78. Il y a quelque chose qui fonctionne, mais ces 3 derniers, donc on va y aller. En fait, nous pensons que nous assistons à un usage répété et amplifié par les forces de l'or depuis quelques années, des bombes lacrymogènes lors des manifestations, voire même lors d'événements sportifs. on connaît les effets sur la santé des des de l'ensemble des personnes qui sont présentes dans la zone où légale sans utiliser de ces gaz, on l'a vu d'ailleurs lors de, de la gestion des incidents du Stade de France l'évacuer 2022, à Saint-Denis, on est bien placé pour le savoir puisque je rappelle pas mais il y a une mission importante du Sénat qui a illustré un certain nombre de problématiques de matières, de l'autre, que nous connaissons aujourd'hui, après avoir entendu en tant que préfet l'Lallement. C'est un mauvais usage pour nous, qui a été dit par exemple démontré à cette occasion, qui avait conduit aussi, alors j'ai pas citer tous les faits divers, mais comme je : je viens de Marseille je vous rappelle quand même cette cette ce fait divers assez dramatique

je vais pas prendre ça pour dire tout va mal, mais simplement pour dire que il y a quand même une utilisation qui nous parler des fois aléatoire ou disproportionné en tout cas, et qui ne paraît pas correspondre à la réalité, en tout cas pour nous de ce qui se passe sur le terrain et en tout cas, porte une vision très très clair d'une forme de Mattel lors très particulière qui nous paraît pas être la seule et qui nous paraît en plus être une attaque quelque part un certain état de droit, donc nous pensons qu'il faut mener une réflexion sur cette doctrine et que nous demandons donc pas cet amendement à ce que le gouvernement dresse un bilan sur l'usage des aérosols lacrymogènes ou incapacitants lors des manifestations et des événements sportifs. Merci, chers collègue monsieur le rapporteur, votre avis. Voilà, président de je pense que la prochaine discussion d'un texte spécifique sur les Jeux olympiques nous permettra de rediscuter la sécurité des événements sportifs et donc l'avis est défavorable à cette demande de rapport. Je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui vote pour, contre, abstention, il n'est pas adopté, nous passons à la le 15, madame la présidente Assassi l'amendement 198. Oui merci madame la présidente, donc cet article 15 renforce le Champ de l'autorité fonctionnelle du préfet sur les services déconcentrés de l'État et les établissements publics, couvrant un large Champ de l'action publique, nous considérons que le régime de l'état d'urgence actuelle permet déjà d'octroyer des prérogatives exorbitantes de droit commun au préfet l'article 15, donc nous semble superfétatoire, il n'est pas nécessaire de la, de l'instaurer spécifiquement dans des zones départementale puisque sur exit ce régime, je le redis existent déjà, d'où l'expression que j'ai utilisé dans la direction discussion générale, à savoir, selon laquelle, pardon, la Lopmi serait l'antichambre de la réforme à venir portant départementalisation de la police judiciaire, donc nous serons. Bien évidemment très avant

c'est un un amendement de suppression de l'article 1 qu'vient de présenter, madame la présidente, cet article qui permet de renforcer les prérogatives des préfets de département en cas d'événements d'une particulière gravité Une autorité sur les services et établissements publics de l'État ayant un Champ territorial et qu'ils sont tous placés sous son autorité, je dirais même, nous avons même a adopté un amendement qui permet même de de placer l'ARS, sous l'autorité du préfet, ce qui est une une bonne chose qui a été votée par la par la commission des lois, donc. je, je ne partage pas les craintes que vous que vous avez évoquées, je crois qu'on a vécu une une période de crise importante, on a d'ailleurs au sénat travailler dès l'année 2020 avec un rapport sur la nation en période de crise sous l'eau le l'empire du de de Philippe Bas à l'époque et je crois que il faut que nous ayons

Merci, c'est donc défavorable, monsieur le Ministre. Parfait, je mets donc aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables qui votent pour, contre, abstention, il n'est pas adopté Monsieur Bénard Roche l'amendement 69. Sur le même article, les sénateurs dans dans le groupe reconnaissent la nécessité de pouvoir assurer au niveau départemental, une dites commandement en temps de crise permettant de garantir la rapidité, l'efficacité, la TJ Villiers l'intelligibilité des décisions à prendre nous considérons que la liste des crises à l'occasion desquelles le préfet est habilité à diriger l'action de l'ensemble des services établissements de l'État est trop large, l'amendement vise donc à recentrer l'habilitation préfectorale pour les événements résultant de la crise climatique qui doivent concentrer toute l'attention de l'appareil d'État le projet inclut en effet ouvrez les guillemets, les événements de nature à entraîner un danger grave et imminente pour la sécurité, l'ordre et la santé publique, formulation qui nous paraît lâche bien trop large et qui permet d'englober par exemple des périodes manifestations de mouvements sociaux d'ampleur et par conséquent de renforcer, à ce moment-là, une certaine forme de réponse de l'État par la main du préfet l'attention disproportionnée que porte le gouvernement sur les menaces à l'ordre public et à la sécurité reflète, me semble-t-il une politique du tout sécuritaire que nous avons dénoncé tout au long de cette loi d'orientation qui n'est bien entendu pas la nôtre puisque nous ne voyons pas leur population une menace potentielle et ne une menace potentielle par ailleurs les auteurs de cet amendement, font remarquer que les menaces sécuritaires et sanitaires font déjà l'objet ou en fait déjà l'objet de régime dérogatoire du droit commun, au travers des états d'urgence sécuritaire et sanitaire et en fait, les auteurs de l'amendement, considère que l'extension des pouvoirs du préfet doit se concentrer sur les menaces climatiques qui vont aller en s'empirant ces prochaines années et décennies il faut d'ailleurs remarquer que l'exposé des motifs du du texte, a dit que, ouvrez les guillemets, tous les scénarios, anticipant les crises de demain convergent vers leur augmentation du fait a minima de phénomènes climatiques extrêmes, ce qui montre bien que l'objet 1er de cette disposition la crise climatique et ses conséquences, feux de forêt épisodes météorologiques extrêmes pénurie de denrées alimentaires alimentaire sécheresse l'été que nous venons collectivement de traverser tempête attends en Corse, feux de forêt dévastateurs doit concentrer toutes les attentions de l'État. Merci, monsieur le rapporteur, à votre avis. Oui je madame la présidente, je ne peux pas partager l'amendement de notre collègue Guy Roche parce que cette, ce travail sur les pouvoirs du préfet, il se fait pour toutes les crises et ne vouloir ne les limiter qu'aux crises environnementales déjà avec ce que ça peut recouvrir de de de question d'interprétation de ce que c'est qu'une crise en grande véranda en tout cas liés au changement climatique, comme vous l'avez comme vous l'avez évoqué non je pense qu'effectivement le préfet dans le département, il doit être le patron des services quand tout va bien, mais il doit être aussi et surtout le patron de tous les services compte là. La, la, la cohésion sociale et et est affecté, évidemment on ne peut pas limiter ça ça seulement aux aux problèmes environnementaux, il y a tous les autres problèmes et au sort d'une crise va en sorte de plusieurs crises, on peut, on peut savoir ce que ça représente, je crois que les préfets encore ces dernières heures ont pris des, des, qui montre que le pouvoir préfectoral dans le département et le pouvoir légitime de l'État, qui représente l'État exécutif et qui doit pouvoir prendre des petites décisions rapides, c'est le bon échelon en tout cas c'est la position de la commission des lois, avis défavorable.

Oui, il s'agit toujours des renforcements de la compétence de torréfier des de l'autorité fonctionnelle du préfet sur les services déconcentrés de l'État, il nous semble qu'il serait utile que les conditions qui préside à cette extension, ce renforcement soient motivés et. Alors et. Alors je je vais madame la présidente, faire part à Jérôme Durain d'une observation que j'ai déjà fait en commission qui ne le surprend le surprendra pas. Vous êtes dans une crise. Importante.

Sur le terrain des crises compliquées, on va pas occupé le les les services de la préfecture de région à s'occuper de ça. Ou alors on risque de tomber sur un quelque chose de, de, de très simple qui est la l'arrêter type, c'est-à-dire qu'on dira, étant donné la gravité de la situation pour 3 petits points et puis, et puis on mettra le nom du préfet de département et puis le on affichera ça la preuve de la porte de la préfecture de région donc honnêtement je, je, j'en comprends l'esprit hein, je ne veux pas du tout remettre en cause le l'idée que vous avez, je pense que sur un plan opérationnel, elle, elle ne revêt non seulement aucun intérêt mais elle alourdit en plus la charge dans une période où, préfet de région, préfet de zone, préfet de région et préfet de département auront entre guillemets, d'autres chats à fouetter, pardon pour cette familiarité que de de s'occuper de produire des arrêtés. Monsieur le Ministre, même avis défavorable. On n'a pas le droit de fouetter les chats, donc je retire ma ma des amendements pour un article additionnel 2 amendements identiques après cet article, Monsieur Durand, l'amendement 42. Un amendement dans le 1er signataire est notre collègue Hussein Bourgi dans son avis du 10 mars 2022 portant sur la première version de la lotte, 1000 Conseil d'État mis en garde sur l'existence d'une certaine érosion des pouvoirs de direction et de contrôle des enquêtes par le parquet, et donc par l'autorité judiciaire, il nous semble, et il semble à l'auteur de l'Arctique, un mécanisme de consultation pour avis pourrait être utilement créée pour que toute réforme à venir, y compris par voie réglementaire concernant l'organisation des services de police ou de gendarmerie en charge de mission de police judiciaire reçoivent la ville simple ou de la Cour de cassation acquis pas acquis applicable, pardon pour la police nationale et la gendarmerie nationale, nous voulons que demeure assurer le principe de la spécificité de services de police nationale et de la gendarmerie nationale dédiée à des missions de police judiciaire, tant à l'échelon national que territorial. Merci monsieur ben Haroche amendements identiques. la police judiciaire doit être placé sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire, le rapport final du comité des états généraux de la justice, a souligné son attachement à ce que la police judiciaire quand il d'exercer directement ses activités sous la direction des magistrats du parquet ou le cas échéant des juges d'instruction, le Conseil d'État, Jérôme Durain, on a parlé vise donc tout d'abord inscrire plus clairement l'exigence constitutionnelle, rappelé par le Conseil constitutionnel dans la partie législative du code de la sécurité intérieure et à lui donner un sens plus concret en fixant des principes fondamentaux pour l'organisation administrative et territoriale des services en charge des missions de police judiciaire au c'est de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et en permettant de prendre en compte l'avis de l'autorité judiciaire sur cette organisation, l'amendement harmonise également les règles applicables pour la police nationale et la gendarmerie nationale, il pose le principe selon lequel doit demeurer, assurer la spécificité des services de police nationale et de la gendarmerie nationale dédié à des missions de police judiciaire, tant à l'échelon national que territorial, enfin, cet amendement vise à garantir le libre choix des officiers de police judiciaire ou des services auquel ils appartiennent, par l'autorité judiciaire compétente, en effet, cette liberté de choix est indispensable pour que l'autorité judiciaire compétente puisse décider selon le contexte, quelles seront les destinataires les plus pertinents de ses instructions ou réquisition l'indépendance des enquêtes judiciaires dépend de ce principe de libre choix des enquêteurs, ça nous apparaît dans 4 poids quand même important, même si c'est pratiquement le dernier de de notre de notre après- midi je préciserai que cet amendement a aussi été proposé par l'Union syndicale des magistrats. Pourtant, votre avis s'il vous plaît. et les assurances que. Le gouvernement tente à nous donner les conséquences pratiques de cette réforme seront examinés par la mission d'information de notre commission des lois, qui a été confié à notre collègue Nadine Bénureau à vous cher Jérôme Durain dès lors, la réaffirmation des principes ne nous semble pas nécessaire à l'échelle de ce texte de loi, par ailleurs, la procédure envisagée pour l'organisation de la police judiciaire paraît particulièrement lourde et complexe avec un avis systématique de la comme Cour de cassation sur un décret qui me semble au contraire à la séparation des pouvoirs, dont l'avis défavorable. Si Monsieur le Ministre, même avis. Je mets donc aux voix ces deux amendements avec 2 avis défavorables qui votent pour, contre, abstention il ne. Sont pas adoptées article 16 madame Conconne vous souhaitez prendre la parole sur cet article. Oui, on arrive à la fin de ce débat et j'ai l'honneur quasiment de le clôturer avec mon amendement, donc on va parler un petit peu de fonds pour qu'on s'en souvienne, hier j'ai eu le bonheur d'de Monsieur le Ministre dire le Sénat n'aime pas les ordonnances, donc j'espère bien que mon amendement à venir sera voté à l'unanimité pour donner du sens à cette déclaration à ce ressenti, c'est toujours comme ça à la fin de texte il y a un petit truc, on rajoute sur l'outre-mer, on va gérer par ordonnance, Monsieur le Ministre, vous savez que vous êtes saisi par plusieurs présidents d'exécutifs, qui souhaite que la donne change dans les relations avec l'État. Vraiment, la donne change et que l'on rentre dans un discours plus démocratique, plus libre, plus construit co-construit Cette redondance d'ordonnance et gênante, je sais que vous partagez mon avis, on en a déjà parlé et vous l'avez dit encore hier, donc, ce serait très bien aujourd'hui de se dire que, compte tenu des problèmes très spécifiques de sécurité que nous avons, plaque tournante de drogue avec des problèmes aux frontières qui sont difficiles à contrôler et qui demande beaucoup de matériel, vous en êtes conscient hier, je vous ai remercié pour les nombreuses décisions que vous avez prise en Live qui sont extrêmement concrètes et pragmatiques et qui devrait donner des résultats très vite, il faut qu'on rentre qu'on ouvre une nouvelle ère de débat avec l'État et que cette cette nouvelle ère, ne soit plus l'abondance d'ordonnances qui nous prive du débat démocratique et que l'on puisse régulièrement pouvoir prévoir des sorties des mentions qui soient spécifiques à des territoires spécifiques et qui soient spécifiques à des situations spécifiques merci. Madame la sénatrice, vous avez parfaitement raison et donc je vous propose que nous votions votre amendement de suppression, je veux dire pourquoi on en est là parce que il y a des comme des dispositions qu'il faut adapter à l'Outre-mer, notamment sur ceux qui disposent de diverses, comment dirais-je, articles de la Constitution différents selon les les territoires ultramarins, est ce que la réponse que m'a faite que mon fait service et qu'une partie de la direction générale qui s'en occupe, nous a pas répondu et il ne vous appartient pas en tant que parlementaire de subir ce que fait mal l'exécutif je propose donc on vote la suppression de l'ordonnance et j'espère que d'ici là ça forcera tout le monde a travaillé pour présenter à l'Assemblée nationale, des dispositions en dur. Merci monsieur le ministre, en attendant, nous avons l'amendement de coordination 232 de la commission des lois, vous mettez un avis favorable. Comme c'est un amendement de coordination, c'est pas très difficile, a présenté monsieur le Ministre, avis favorable je fais donc voter cet avis. Favorable sur le 232 ceux qui votent pour, contre, abstention il était adopté, l'amendement 52 madame Conconne vous venez de le présenter, il a un avis favorable du gouvernement, la commission.

Madame Conconne pour explication de vote. Explications de vote, je ne peux que saluer cette décision unanime du Sénat supporter aussi bien par la commission que par le ministre de l'Intérieur, je pense qu'aujourd'hui on ouvre une nouvelle ère. Monsieur : Théophile pour explication de vote.

l'avis du ministre et et l'approbation de l'Assemblée, encore une fois les on a bien compris, vous avez bien compris la difficulté, je pense que les récentes crises nous ont permis, tout ça nous tous de de comprendre qu'il y a véritablement un enjeu là et que nous pouvons répondre à des préoccupations au travers nos, nos discussions. Qui vote contre, c'est une belle unanimité, bravo, merci, Monsieur le Ministre, je mets au vote, l'article 16 ainsi modifiée avec qui vote pour qui votent contre, qui s'abstient, il était adopté, nous avons donc terminé l'examen des articles de ce texte, je vous rappelle que les et puis, explications de vote et le vote par scrutin public solennel. Sur l'ensemble du projet de loi se dérouleront le mardi 18 octobre à 14 heures 30 nous vous y attendons Monsieur le Ministre, mais en attendant, je pense que vous voulez avoir un mot de conclusion. Ce qu'on a la présidente pour vous remercier, remercier Monsieur le Président commission d'rapporteur, et je pense ensemble des des orateurs pour ce texte qui est important, j'espère que tout le monde aura compris l'esprit dans lequel est venu le gouvernement dire et remercié la commission des lois pour son travail, que nous a éclairés, je crois qu'on a pris en compte ces sujets et terminaient pas dire la sénatrice con que je suis très sensible à l'argument qu'à la fin il y a toujours l'outre-mer, ont fait une ordonnance, on parle pas tellement des sujets et vous avez effectivement le droit de parler de tous les sujets ultra-barrages sont très important, sans doute, et tu sais une amélioration, que le ministre de l'Intérieur soit aussi outre-mer pour avoir ce genre d'argument merci. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre, je vais lever la séance prochaine séance mardi 18 octobre à 14 heures 30 pour ces explications de vote, la séance est levée, bonne soirée.